Sept minutes ont suffi pour plonger la préfecture de police dans l'un des drames les plus douloureux de son histoire et la France dans l'incompréhension et la stupeur. » Les mots du Président de la République ont été forts. Ils ont été justes. Au nom des sénateurs du groupe La République En Marche et de tous mes collègues, je souhaite me joindre à la solidarité unanimement exprimée à l'égard des familles, des victimes et de l'ensemble des forces de l'ordre. Le 3 octobre dernier, la France a été frappée au coeur du symbole de l'ordre républicain. L'heure est à la peine et à la douleur. Nul doute que l'enquête judiciaire permettra de faire toute la lumière sur les circonstances de cet acte et sur les motivations de son auteur. Mes chers collègues, nous devons faire bloc. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais saluer le travail des services de renseignement, qui, quotidiennement, déjouent nombre d'attentats, et ce aux quatre coins de l'hexagone- 59 attentats ont été déjoués depuis 2013. Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé combien l'État entend lutter avec force et détermination contre les dysfonctionnements éventuels dans l'ensemble de nos institutions. Sachons traquer la radicalisation partout, au coeur des services de l'État, dans nos écoles, nos transports ou nos hôpitaux. Pour ce faire,

sur les éventuels signalements, l'autre sur l'ensemble des services de renseignement spécialement impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous évoquer les pistes sur lesquelles vous travaillez pour prévenir les dérives et les dysfonctionnements potentiels, dans ce domaine ô combien difficile ? La parole

à telle époque ou dans tel service, n'aurait pas été à la hauteur des enjeux. Je veux le dire très simplement très sincèrement : à partir de 2015, les gouvernements qui se sont succédé ont fait de leur mieux pour parer aux urgences les plus pressées et éviter dans la mesure du possible la commission de nouveaux attentats.

les services de renseignement et les forces de l'ordre, qui remportent semaine après semaine des victoires face au terrorisme. Leurs victoires sont toujours discrètes, et parfois nous n'en parlons même pas, mais elles sont réelles, tandis que leurs échecs sont toujours spectaculaires et dramatiques.

Non-partage de la valeur, aléas climatiques et sanitaires, lourdeurs administratives, CETA et, maintenant, zone de non-traitement. Hier, les agriculteurs ont crié leur détresse. Cessons de tirer sur l'ambulance ! Un agriculteur se suicide tous les jours. Cela ne suffit-il pas ? Que veut cette société qui se clive dangereusement ? Faire disparaitre notre agriculture ? S'alimenter avec des produits importés qui ne respectent pas nos propres exigences sanitaires ? Pourquoi accuser inlassablement nos agriculteurs ? Je rappelle qu'ils n'utilisent que des produits homologués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, seule légitime pour les autorisations de mise sur le marché. Il n'y aura pas de transition écologique sans nos paysans. Ils l'ont compris et veulent y jouer un rôle fondamental et répondre à l'attente sociétale. Pourquoi ne parle-t-on pas de tous les efforts entrepris depuis des années pour s'inscrire dans une agriculture durable ? Pourquoi ne cibler que le mauvais, sans jamais parler du bon ? Le bon, c'est par exemple VitiREV, un

Il faut agir collectivement, selon une véritable stratégie coconstruite avec la filière, les consommateurs, les distributeurs et les industriels, en traçant une ligne unifiée et partagée. Monsieur le ministre, personne ne peut nier votre soutien aux agriculteurs : votre combat contre l'agri-bashing est constant. Mais quelle est la cohérence quand l'État encourage une transition agroécologique et que, en même temps, il vide les chambres d'agriculture de leur contenu et de leur proximité dans une simple logique budgétaire ? Ce projet ambitieux ne réussira pas sans les chambres d'agriculture

l'alimentation fournie par nos agriculteurs est la plus sûre, la plus saine et la plus durable d'Europe. Monsieur Cabanel, vous avez raison, ce dénigrement, cet agri-bashing, est totalement insupportable,

Pour autant, aujourd'hui, des chars et des véhicules blindés se dirigent vers la frontière ; une offensive est imminente. Pour les Kurdes, cette zone de sécurité équivaut à une zone de péril et de mort certaine. États-Unis ou pas, de toute façon, Erdogan se moque totalement du droit international et s'allie sans vergogne avec des mouvements islamistes contre les Kurdes. Pourquoi se priverait-il ? À chaque nouvelle offensive, aucune sanction réelle de la communauté internationale ! L'abandon programmé des Kurdes syriens ne constitue pas seulement une faute morale ; c'est aussi une faute stratégique. Rappelons-nous bien que, si l'État islamique n'existe plus aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux combattants et combattantes kurdes- je pense notamment à ces femmes formidables. Faut-il désespérer de l'influence de notre gouvernement dans ce conflit ?

Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, voilà quelques jours, plus de 20 000 policiers manifestaient pour exprimer leur malaise. La crise dans la fonction publique hospitalière est telle que Mme la ministre des solidarités et de la santé reconnaît elle-même que le pacte de refondation des urgences sera insuffisant pour calmer les esprits. Médecins, infirmiers, pompiers sont tous exposés, en première ligne, à la précarité, aux violences de la société. Les drames récents dans l'éducation nationale illustrent également ce désespoir lié à l'absence de reconnaissance en l'occurrence des personnels enseignants. Dans ce contexte de défiance, la réforme territoriale de la direction des finances publiques, menée au pas de charge, vise en réalité à supprimer plus de 2 000 postes dès l'année prochaine, et 15 000 à terme. Monsieur le ministre, personne n'est dupe : derrière l'annonce de cette réforme se dissimule un nouveau transfert de charges vers les collectivités territoriales. Or, vous le savez pertinemment, les dotations financières de l'État pour le fonctionnement des maisons France services seront largement insuffisantes. Les seuls interlocuteurs de nos concitoyens seront des animateurs généralistes dont ne nous savons rien aujourd'hui de leur formation ou de leurs compétences. Avec cette privatisation déguisée du service public, vous n'offrez aucune garantie, et notamment celle de la confidentialité, surtout quand ces tâches sont confiées à des buralistes, de moins en moins nombreux dans un monde rural une nouvelle fois

assument, sans moyens affectés, le rôle d'écrivain public et numérique. Monsieur le ministre, quels sont vos objectifs de réduction d'effectifs et de maintien des services publics de proximité ? Quelles garanties nous apportez-vous ? Comment repensez-vous le rôle des communes et des EPCI, qui devront pallier les difficultés d'accessibilité numérique ?

l'impôt à la source, souhaité notamment par votre groupe politique, voilà quelques mois encore, la déclaration tacite du revenu à partir de l'année prochaine et la suppression de la taxe d'habitation. Je rappelle que 4 000 agents

président. Monsieur le ministre, je crains simplement que ces mesures ne continuent à creuser la fracture territoriale, à renforcer l'insécurité financière et juridique des citoyens et des élus locaux, surtout ceux qui sont éloignés des centres de décision. C'est en total contresens avec les attentes actuelles

Monsieur le ministre, les 15 et 22 mars prochains, les Français vont vivre un moment de démocratie très important en renouvelant, sur tout le territoire, les conseils municipaux de chacune de nos villes, de nos communes, de chacun de nos villages. Cette période électorale approchant, de nombreux maires indépendants, sans étiquette et non-inscrits, m'ont interrogé au sujet de la nuance politique qui leur sera attribuée par l'administration. En effet, c'est le ministère de l'intérieur qui procède à l'attribution de nuances politiques dans un cadre strictement défini juridiquement,

portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel, a confirmé tout l'intérêt de l'attribution de ces nuances. Lors du dépôt de candidature, le candidat déclare s'il se présente avec une étiquette politique ; il peut aussi se déclarer « sans étiquette » ou « indépendant Ce sont alors les préfets- loin de moi l'idée de remettre en cause leur don de discernement -qui attribuent la nuance sur les critères suivants : connaissance historique des candidats ; programme du candidat ; investiture ou soutien reçu. Pour les communes de 1 000 habitants et plus, c'est avant le scrutin ; pour les communes de moins de 1 000 habitants, c'est après l'élection du maire. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, si vous souhaitez intégrer dans la grille des nuances politiques les classifications « sans étiquette

3 500 ou 9 000 habitants, en deçà duquel l'appartenance politique aux grands courants que nous connaissons n'est pas indispensable. Je suis, sur ce sujet, totalement à votre écoute.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, j'aurais aimé ne pas avoir à reprendre la parole dans cet hémicycle après une nouvelle frappe de l'islam radical. Malheureusement, l'histoire bégaie. Après Paris, Nice,

aux quatre policiers lâchement assassinés, à leurs familles et à l'ensemble de leurs collègues endeuillés. Le Président de la République parle de bâtir une société de vigilance. Est-ce à dire qu'il entend exonérer sa propre responsabilité et qu'il veut faire porter injustement une part de responsabilité aux Français ? N'importe quoi ! Or ce qui s'est passé à la préfecture de police d'une longue dégradation, de compromis et de la chape de plomb que fait peser dans l'espace public le politiquement correct. Ce n'est pas en jetant à la figure de ceux qui s'inquiètent du désarmement moral de notre société et de sa communautarisation le qualificatif « islamophobe

Vos mots ne suffiront plus, et ce sont vos actes, désormais, qui seront jugés. Monsieur le Premier ministre, allez-vous vraiment vous attaquer au terreau de l'islamisme et à toutes les formes de communautarisme ?

un risque. Plus globalement, il n'y a pas un jour, pas une heure, où nos services ne sont pas mobilisés pour déjouer un risque, pour qu'un risque éventuel ne devienne pas un risque avéré. M. le Premier ministre a rappelé les 59 attentats terroristes qui ont été neutralisés grâce à l'intervention de nos forces de sécurité intérieure. Mais nous devons effectivement être extrêmement vigilants pour ne rien laisser passer qui soit une atteinte à la République et une menace pour les Français. Je vais être très factuel, madame la sénatrice, pour vous donner quelques indications

des paroles aux actes ! Vous le savez très bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à vous défausser sur la société. L'État, lui seul, doit prendre toutes ses responsabilités,

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, les paysans étaient hier dans la rue. Ils sont dans une situation difficile et multifactorielle dont ils ne voient pas l'issue.

On leur demande d'être exemplaires, sans craindre des concurrents qui le seraient moins ; on leur demande de nous nourrir, et on les suspecte de nous empoisonner. Et maintenant, cette terrible sécheresse achève de les mener au désespoir. De nouveau, des forces contradictoires se manifestent. D'un côté, il y a vous, monsieur le ministre de l'agriculture, que j'ai entendu dire

aucune différence, aucune divergence entre le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la simple

Non, on ne peut pas regarder l'eau tomber du ciel pendant six mois, et la chercher les six autres mois de l'année. On sait très bien que le réchauffement climatique va continuer et que, si nous voulons que l'agriculture française soit résiliente, il faudra qu'elle soit irriguée.

Je veux tout d'abord m'incliner devant la douleur des familles, leur exprimer ma solidarité et saluer, au nom de mes collègues sénateurs, le sacrifice des victimes : Aurélia Trifiro, Damien Ernest, Anthony Lancelot, Brice Le Mescam. Permettez-moi d'avoir moi aussi une pensée pour nos amis allemands, victimes de l'attaque d'une synagogue. Monsieur le ministre, j'aimerais que nous puissions nous en tenir aux faits et comprendre ce drame gravissime. Depuis 2015, des dizaines d'attentats ont été déjoués grâce aux services de renseignement. Je souhaite saluer le travail de nos forces de l'ordre. Mais comment un membre de ces services a-t-il pu prendre pour cible ses camarades ? Comment un terroriste a-t-il pu travailler dans un lieu dont la mission est d'identifier les individus dangereux ? Cet attentat implique de surcroît un informaticien qui disposait de l'accès à un nombre important d'informations sensibles. À quels fichiers pouvait-il accéder ? Avez-vous identifié ses contacts en France et à l'étranger ? Quelle protection est mise en oeuvre pour les policiers potentiellement en danger ?

N'aurait-il pas été plus prudent de vous en tenir à la compassion et au constat de la gravité de la situation ? Le phénomène de radicalisation existe au sein de l'administration dans des secteurs stratégiques. Nous devons être capables d'écarter ces personnes radicalisées et porteuses d'une idéologie claire : détruire notre société démocratique et les valeurs qu'elle représente. Enfin, monsieur le ministre, je vous invite, pour terminer, à un peu d'introspection quel phénomène de cécité, de faiblesse, de lâcheté ou de crainte a-t-il pu conduire à l'absence de réaction ? La parole

va diligenter une enquête auprès de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris pour essayer de comprendre pourquoi ces signaux n'ont pas abouti à un signalement, ce qui, je vous le concède, peut paraître extrêmement aberrant dans un service chargé de la lutte antiterroriste. C'est tout cela qu'il nous faudra élucider.

qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. « L'offre de soins est en train de se renforcer et les Français le voient », déclarait Mme la ministre il y a moins d'un mois. Sans vouloir gâcher cet optimisme, je souhaite attirer son attention sur la situation catastrophique de nos services d'urgence. Un peu partout en France, depuis six mois, nous constatons tous la recrudescence de dysfonctionnements à répétition dans les services d'urgences hospitalières. Tel est le cas dans mon département, la Sarthe, à l'hôpital du Bailleul. L'année dernière, j'avais alerté, à propos de cet établissement, sur l'accès à l'IVG, en raison d'un manque de médecins. et de réanimation, ou SMUR, qui est à l'arrêt, faute de médecins urgentistes ! Véritable hôpital de proximité, le Pôle santé Sarthe et Loir dessert un bassin de vie de plus de 150 000 habitants dans un territoire rural. Une réorganisation des personnels ne réglera pas cette dégradation constante de l'offre de soins, qui ne cesse de s'aggraver, la aussi bien dans la Sarthe que dans l'ensemble du territoire français. En revanche, les personnels lui demandent, depuis des mois, des mesures très concrètes en termes de lits, de recrutements, de revalorisations salariales, ou encore de moyens supplémentaires.

Après la désertification médicale, nous arrivons à un nouveau stade de la décomposition du paysage sanitaire. Face à un maillage qui craque, les mesures proposées ne répondent pas à l'anxiété grandissante des populations, qui voient leurs services d'urgence fermer un à un-

par l'agence régionale de santé, l'ARS, et par les autres hôpitaux du groupement hospitalier de territoire. Il est apparu pour l'instant impossible d'avoir un médecin disponible pour assurer son service la nuit dans cet hôpital. Or cette présence, vous en conviendrez, madame la sénatrice, est indispensable pour garantir la sécurité des patients. Dans l'attente, nous avons souhaité que les urgences puissent rester ouvertes la journée, avec la présence d'un médecin, et que la nuit, une infirmière et une aide-soignante soient en mesure d'orienter les patients, évidemment en lien avec la plateforme du 15. Vous le savez, la ministre a eu l'occasion de présenter un plan d'action pour les urgences, qui est doté à hauteur de 750 millions d'euros. Ce n'est pas assez ! Ce plan permettra de réaliser des recrutements en nombre.

pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Nous ne pouvons naturellement nous satisfaire de la réponse qui vient d'être faite à notre collègue Lons-le-Saunier, fermeture de la deuxième ligne du SMUR ; Ploërmel, fermeture du SMUR cet été ; Sisteron, fermeture des urgences de nuit depuis le mois de juillet ; Lens, fermeture partielle des urgences cet été ; Toulouse, fermeture temporaire des urgences de nuit ; Mulhouse-Sud-Alsace, fermeture temporaire des urgences : je pourrais encore poursuivre

25 000 personnes qui se présentent chaque année aux urgences de cet établissement, lequel dessert un bassin de population de 150 000 habitants et où il manque neuf médecins urgentistes. Plus généralement, c'est donc la double peine pour les territoires ruraux, leurs médecins généralistes qui partent en retraite ne sont pas remplacés et les services d'urgence de leurs hôpitaux ferment. Dans de nombreux départements, lorsque les urgences ne sont pas fermées par manque de médecins urgentistes, leur personnel est en grève La réponse gouvernementale n'est pas à la hauteur des attentes des professionnels de la santé et des territoires. Aujourd'hui, les personnels sont au bord de l'épuisement. Que compte faire Mme la ministre pour juguler ce mouvement qui s'amplifie ? Que compte-t-elle faire, face à la pénurie de médecins urgentistes dans nos hôpitaux ?

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce gouvernement a réalisé, en matière de santé, des efforts considérables. Je veux vous rappeler quelques faits. Depuis dix ans, nous sommes, le premier gouvernement à avoir augmenté les tarifs hospitaliers, à avoir restitué aux hôpitaux la totalité des crédits qui ont été mis en réserve.

assurer ainsi un meilleur service à la population. Dans les trois ans qui viennent, ces mesures vont être portées à 750 millions d'euros. D'ores et déjà, conformément aux premières annonces faites par la ministre des solidarités et de la santé, les personnels soignants des urgences ont vu apparaître, cet été, sur leur fiche de paye, une prime de risque d'un montant de 100 euros nets, sans compter la prime de coopération qui leur sera attribuée. De manière générale,

La difficulté, c'est aussi le recrutement. C'est la raison pour laquelle nous avons fait sauter le verrou du, ... Ce n'est pas vrai ! ... qui, depuis bien longtemps, pose problème dans notre pays. Nous ouvrons des lits post-urgences lorsque c'est nécessaire. Une transformation en profondeur est engagée. Soyez assuré que nous allons la poursuivre. Pierre Vogel, pour la réplique. La crise des services d'urgence est sans précédent ! Nous sommes à un point de rupture, mais à l'évidence, le Gouvernement ne mesure pas le niveau d'alerte. Vos propositions ne répondent en rien aux besoins des professionnels de santé et des populations, madame la secrétaire d'État. Pis, la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dévoile un plan d'économies de plus de 4 milliards d'euros, qui touchera encore le secteur de la santé. Dans ce tableau déjà sombre, ce sont les établissements de santé qui seront les moins bien lotis. Ce sont donc encore les personnels hospitaliers, les patients qui devront supporter les conséquences de ces économies, avec tout ce que cela implique en termes de prise en charge du malade auquel vous faites prendre des risques inconsidérés.

Plusieurs effets se conjuguent : sécheresses à répétition, fortes chaleurs, attaques parasitaires, dégâts de gibiers croissants ... Aujourd'hui, plus aucune essence, plus aucun territoire n'est épargné. À ce stade, les dégâts dans les grandes régions forestières se chiffrent à plus de 2 millions de mètres cubes. On prévoit 5 à 6 millions- soit plusieurs années de récoltes -au printemps prochain, car beaucoup d'arbres ne repartiront pas. À la catastrophe écologique s'ajoute le désastre économique : des communes forestières privées de recettes, des marchés saturés, des prix qui chutent et, demain, des trous de production qui ne permettront plus d'alimenter les besoins en constructions ou en charpentes. Le risque incendie s'intensifie lui aussi et se répand, menaçant des régions situées beaucoup plus au nord. Face à ces réalités liées au changement climatique qui s'accélère, il nous faut, dès à présent, adapter nos forêts : privilégier des essences plus résistantes, plus sobres en eau, diversifier et mélanger nos essences.

productrice de bois d'oeuvre et de puits de carbone. Le Gouvernement français tarde à s'emparer de ce sujet. Voilà des mois que les forestiers tentent de récolter et de transformer les arbres qui peuvent encore l'être. C'est une course contre la montre pour essayer d'endiguer la propagation des parasites, chercher des débouchés.

pour regarder ce que va devenir la forêt française dans les années à venir. Oui, nous examinons ce qui se passe dans cette forêt ! Il y a deux problèmes, que vous connaissez bien mieux que moi, madame la sénatrice. D'abord, le problème parasitaire, avec les scolytes, auquel nous essayons de répondre. Nous venons de mettre 16 millions d'euros en argent sonnant et trébuchant sur la table

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, le 21 septembre dernier, dans le huis clos de son école vide, à Pantin, une directrice se donnait la mort. Elle s'appelait Christine Renon. Elle avait cinquante-huit ans. Le même jour, à Nice, à son domicile, professeur de biologie disait adieu à la vie. Il s'appelait Frédéric Boulé. Il avait, lui aussi, cinquante-huit ans. Chaque semaine, la liste des fonctionnaires qui se suicident s'allonge : policiers, enseignants. Ils se suicident parce qu'ils sont à bout, épuisés ; parce qu'ils se sentent de moins en moins considérés ; parce qu'ils sont mal payés ; parce qu'ils sont parfois insultés, agressés ; parce qu'ils sont stigmatisés, enfin, alors qu'ils sont tout sauf des privilégiés, comme nos amis agriculteurs. Si chaque suicide garde une part de mystère, Christine Renon n'est pas partie dans le silence : elle a laissé une lettre à ses collègues, un appel à ouvrir les yeux. Je n'en lirai qu'une phrase : « Je dois dire aussi que je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous apporter notre institution. » Depuis des années, dans l'éducation nationale, les réformes se succèdent, s'accumulent. Pourtant, le malaise persiste et même empire. La confiance dont parlait Christine Renon et qui ornait le titre de votre loi, monsieur le ministre, est rompue. Je sais votre attachement aux professeurs. Mais que répondez-vous à ces directeurs et enseignants en souffrance, se plaignent de ne pas être écoutés et de voir toutes ces réformes élaborées sans leur accord, tandis que l'école est le réceptacle de tous les maux de la société

Ne nions pas la souffrance qui s'exprime dans le monde enseignant ! Ce que demandent directeurs et enseignants, monsieur le ministre, c'est d'être mieux protégés et soutenus lorsque leur autorité est contestée par certains parents et élèves. C'est aussi d'être mieux payés

harcèle sans plus les comprendre ! Ce mal-être de notre école n'est pas anecdotique. Si nos enseignants ne sont plus les hussards noirs conquérants du temps de Jules Ferry, ils demeurent les piliers de la République. Lorsqu'ils vacillent, c'est la France qui est en danger

chaque semaine, de manière exemplaire et pacifique, dans les plus petits villages comme dans les grandes villes, pour conquérir sa liberté. Si personne ne demande à la France d'agir en lieu et place de la société algérienne, le silence du Gouvernement sur ces événements est chaque jour plus gênant. Depuis quelques semaines, un nouveau cap a été franchi par la junte au pouvoir : on relève des arrestations arbitraires et l'incarcération de citoyens algériens qui expriment simplement leur opinion.

notamment en matière de lutte contre le terrorisme ; pour autant, ne laissons pas le cynisme politique l'emporter sur l'honneur de notre pays ! Il est temps de condamner clairement les agissements contre le mouvement démocratique. À la faute morale, n'ajoutons pas une faute politique N'oublions jamais que c'est le peuple algérien qui est notre allié, et non la junte en place. Il faut tendre la main au peuple algérien : voilà l'intérêt de la France ! C'est bien le peuple algérien qui sera au pouvoir, tôt ou tard : c'est inéluctable. C'est lui notre partenaire, c'est lui l'avenir ! Ne passons pas du silence gêné au silence coupable ! Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple : le Gouvernement compte-t-il condamner les arrestations et les incarcérations d'opposants politiques en Algérie ?

le 9 juillet dernier. Deux voies parallèles continuent de coexister : celle des manifestants, qui expriment une aspiration forte et profonde à ouvrir un nouveau chapitre de l'Algérie, et celle des autorités, qui repose sur la volonté de faire en sorte que la Constitution algérienne puisse s'appliquer en l'état. ? Dans ce contexte, le seul souhait de la France est que les Algériens trouvent ensemble les chemins d'une transition démocratique. C'est ce que nous espérons pour l'Algérie, compte tenu de la densité et de la profondeur

Nous avons confiance dans l'esprit de responsabilité, de civisme et de dignité qui prévaut depuis le début des manifestations et qui suscite l'admiration. Nous sommes attentifs à ce que cet esprit puisse continuer à s'exprimer pacifiquement, dans le respect de la liberté d'expression et de manifestation. Il n'y a qu'une solution : le dialogue démocratique. Nous continuerons à nous tenir aux côtés de l'Algérie et des Algériens, dans le respect et l'amitié qui président à nos relations.

ces opposants, ces citoyens algériens, puissent être libérés ? Ils sont aujourd'hui en prison sans aucune raison. Il faut conclure ! Je compte recevoir une réponse un peu plus précise que celle que vous venez de nous donner.

Au regard du temps long et des enjeux que nos sociétés doivent relever aujourd'hui dans l'urgence, le malaise qu'éprouvent les agriculteurs s'inscrit en réalité dans une crise de civilisation. Nous devons tous, collectivement, faire évoluer nos paradigmes, dans l'agriculture, bien sûr, mais aussi dans les transports, le logement, ou encore l'énergie. S'il y a malaise dans la civilisation- j'estime qu'à bien des égards nous en sommes là -, les agriculteurs ne doivent pas être les boucs émissaires d'une problématique qui concerne en réalité l'entière communauté des citoyens. Les paysans ne sont pas le problème : ils sont l'une des solutions aux difficultés que nous devons résoudre collectivement et dans l'urgence. Alors, monsieur le ministre, au vu de ce contexte, quelle est votre stratégie, quel est votre plan d'action ? Où en êtes-vous de la mise en place des prestations pour services environnementaux, ou PSE, qui permettraient que soit reconnu ce qu'apportent les agriculteurs à la société dans son ensemble, au-delà des biens nourriciers ? Comment allez-vous compenser la baisse des crédits de la politique agricole commune pour la transition vers le bio, ou pour la compensation des handicaps naturels ? Qu'envisagez-vous de faire pour la réalisation rapide d'ouvrages hydrauliques ?

des agriculteurs de France.

En Normandie et en Picardie, plus de 900 exploitations agricoles sont à l'arrêt. Près de 700 000 litres de lait sont détruits chaque jour, pour un manque à gagner déjà supérieur à 3 millions d'euros. Les agriculteurs attendent avec impatience et appréhension les résultats des analyses des suies retombées sur les sols. Vous les annoncez pour la fin de semaine, mais pour eux, chaque jour qui passe est un jour de trop ! Plus grave encore, à ce jour, pas un centime ne leur a été versé. Vous comptez faire payer le pollueur, mais en attendant, c'est à la solidarité nationale de prendre le relais.

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence, dans la tribune d'honneur, d'une délégation du groupe d'amitié de l'Assemblée de la République de Macédoine du Nord, conduite par le président du groupe d'amitié, M. Ivanov. Cette délégation est reçue au Sénat par le groupe interparlementaire d'amitié France-Balkans occidentaux,

avec le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Christian Cambon. Mes chers

L'ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique migratoire de la France et de l'Europe,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs,

qui a sans doute ses limites, mais qui est, je le crois, profondément utile. L'exercice est difficile, parce que, nous le savons, les questions migratoires suscitent plus facilement l'affrontement que le consensus.

sur la nécessité d'« assurer le triomphe de la conception républicaine, ouverte, de la Nation, celle qui assure des droits pour chacun et fait accepter des devoirs pour tous.

Je ne doute pas que si nous avions annoncé ces détails, on nous aurait dit que le débat était faussé et ne servait à rien. Mesdames, messieurs

où une simple phrase ou expression formulée par un des participants, sans jamais avoir besoin d'insister sur ce qu'elle pouvait impliquer, était immédiatement comprise, reçue et partagée par l'ensemble de l'assistance comme un non-dit, mais un non-dit qui aurait fait consensus.

Je ne suis pas sûr que cette situation soit plus favorable ou plus bénéfique que le fait d'avoir un débat explicite, public, devant la représentation nationale.

Il est très facile, je crois, de tourner presque à vide sur le sujet de l'immigration, en ressassant les mêmes obsessions, comme le fantasme du grand remplacement ou l'appel généreux et général à ouvrir grand nos frontières. Il est beaucoup plus difficile de congédier toute forme de facilités ou de rhétoriques pour essayer d'agir avec sagesse et bon sens. C'est ce que méritent évidemment nos concitoyens. Et c'est, je le crois, l'unique manière de bâtir une nation et une Europe fortes, solidaires et crédibles, qui resteront solidaires et crédibles, qui resteront attractives sans être débordées ni repliées sur elles-mêmes. La politique migratoire que nous présentons et sur laquelle nous souhaitons réfléchir avec le Sénat Sénat doit d'abord s'inscrire dans le contexte mondial et européen d'aujourd'hui. Mener une politique d'immigration cohérente n'est pas seulement une affaire de procédures franco-françaises. Il s'agit,

J'évoquerai par exemple l'augmentation de 60 % du nombre de laissez-passer consulaires obtenus dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Tous ceux qui connaissent le sujet le savent, le nombre de laissez-passer consulaires demandés par l'administration française était faible,

Au-delà de cette relation diplomatique forte avec les pays d'origine, je suis convaincu que l'aide publique au développement, pour laquelle nous consentons des efforts financiers croissants- amenés à progresser avec le temps -, doit être mobilisée au service de notre stratégie migratoire. Oui, cela doit s'inscrire dans une relation d'engagements réciproques avec nos partenaires Cette approche sera déclinée dans le projet de loi de finances dont vous débattrez bientôt. Elle donnera lieu aussi à un projet de loi de programmation et d'orientation en matière de développement ; nous vous proposerons de l'examiner au cours de l'année 2020. C'est là la première orientation de la stratégie que vous propose le Gouvernement. La question est souvent discutée, parfois contestée. À nos yeux, il faut assumer de faire de l'aide publique au développement

Dans ce contexte mondial, la situation de l'Europe est particulière. Nous ne sommes plus au coeur de la crise des réfugiés des années 2015 et 2016. Mais les problèmes restent là ; ils sont parfois entiers. Nous avons construit l'Europe de la libre circulation : c'est bien. Nous devons aujourd'hui construire l'Europe de la protection des frontières extérieures : c'est urgent ! Et à l'intérieur de l'Europe, nous devons traiter le problème des mouvements secondaires, qui sont le symptôme et parfois la conséquence d'une gestion encore insuffisamment coordonnée entre les États. Dès que la nouvelle Commission européenne sera installée, le 1 novembre prochain, nous ferons valoir nos propositions de renforcement juridique et opérationnel de la protection des frontières extérieures, et de réforme du régime d'asile européen. Nous veillerons à un bon équilibre entre responsabilité et solidarité pour la gestion des mouvements migratoires à l'intérieur de l'Europe. C'est le deuxième axe nécessaire de nos travaux. Nos concitoyens veulent aussi que nous soyons capables de mieux accueillir et de mieux intégrer. Mieux accueillir, c'est d'abord réduire des délais d'instruction des demandes d'asile qui sont bien trop longs.

Alors que le nombre de demandes d'asile est en très forte augmentation, ces efforts constants ont permis de stabiliser les délais. Mais nous ne sommes pas dans le raccourcissement des délais que nous souhaitions : ce que nous avons gagné à l'instruction, nous l'avons perdu au contentieux. Pour le dire en termes un peu crus, l'instruction est plus rapide qu'auparavant, mais le contentieux des mesures prises a eu tendance à s'allonger, en raison à la fois d'un mouvement de grève qui a frappé la Cour nationale du droit d'asile et d'un

Mieux accueillir consiste surtout à mieux intégrer ceux qui ont vocation à rester. Nous avons déjà fait beaucoup, en donnant une nouvelle ambition au contrat d'intégration républicaine, qui repose désormais sur trois piliers : la langue française, le travail et les valeurs républicaines. nous avons doublé le volume horaire des cours destinés aux primo-arrivants qui en ont besoin. Le respect de nos valeurs républicaines n'est pas non plus négociable, par exemple quand il s'agit de laïcité ou du droit des femmes.

Elles sont dans notre conception universelle : elles ont vocation à s'appliquer universellement. Mais elles ne sont pas toujours partagées,

Cohen nous raconte qu'il avait même érigé un petit autel à la France, avec des figures aussi diverses que Victor Hugo, Jeanne d'Arc ou Napoléon. Je n'en demande pas tant à ceux qui arrivent aujourd'hui, quoique s'ils veulent apprendre par coeur, ce sera toujours bienvenu ! En revanche, nous leur demandons, et nous n'avons pas d'autre choix que de leur demander d'adhérer aux valeurs qui ont fait la France. C'est la raison pour laquelle nous avons modernisé et doublé la durée de la formation civique. Nous devons être inflexibles sur cette exigence. Nous le savons, aucune intégration ne saurait être durable et réussie sans accès au monde du travail. C'est là notre quatrième axe : l'intégration par le travail. Nous avons ajouté un volet « insertion professionnelle » au contrat d'intégration républicaine. républicaine. Nous avons déjà réduit de neuf mois à six mois le délai au terme duquel les demandeurs d'asile peuvent accéder au marché du travail. Et nous soutenons de très nombreux projets d'intégration par l'emploi. Comme souvent, les initiatives qui apportent des solutions émanent de nos territoires ; elles nous ouvrent la voie, mais elles ne suffisent pas. Il faut donc faire plus et mieux. Les procédures d'accès des étrangers au monde du travail doivent être plus globalement repensées. Je propose que nous réinventions le système d'autorisation de travail pour les métiers en tension. La révision de cette liste devrait ainsi permettre de mieux intégrer les étrangers présents en France et d'attirer, lorsque c'est nécessaire, les talents dont notre pays a besoin. Mieux accueillir, c'est aussi assumer un pilotage par objectifs de l'admission au séjour. Nous savons que la logique des quotas ne peut s'appliquer ni en matière d'asile ni en matière d'immigration familiale. Mais, pour attirer les talents, qu'il s'agisse d'étudiants, de compétences rares, ou de compétences dont nous avons besoin, on doit pouvoir réfléchir à des objectifs quantitatifs. C'est là notre cinquième orientation. On doit pouvoir adapter et dynamiser nos procédures d'immigration professionnelle en fonction des besoins des secteurs d'activité. On doit pouvoir se fixer des objectifs en nombre d'étudiants accueillis, en nombre de « passeports talents » délivrés, ou encore sur la proportion de l'immigration qualifiée au sein de l'immigration professionnelle. Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne doit pas y avoir d'angle mort dans notre débat. L'accès à la nationalité ne doit pas être un angle mort. J'ai déjà affirmé lundi, et je la redis aujourd'hui à cette tribune, mon opposition à la suppression du droit du sol. Mais je suis favorable à ce que nous élevions les critères de naturalisation par décret, notamment en ce qui concerne le niveau de maîtrise de la langue française. Nous irons dans cette direction. Il n'y a pas de tabou non plus sur l'immigration familiale : nous lutterons fermement contre les fraudes et les abus. Nous pouvons et nous devons resserrer les critères là où cela se révèle nécessaire. Mesdames, messieurs les sénateurs, pour bien accueillir, il faut se donner les moyens d'une meilleure maîtrise des flux migratoires. Nous devons d'abord comprendre pourquoi le système français d'asile est actuellement saturé. Les mouvements migratoires secondaires expliquent une part importante de la situation. En 2018, 30 % des demandeurs d'asile en France avaient déjà déposé une demande dans un autre État membre, et ne relevaient donc pas de la responsabilité de notre pays. Et beaucoup de ces demandeurs sont issus de pays que l'Ofpra considère comme sûrs. Il y a probablement plusieurs déterminants à ces phénomènes. Mais nous devons regarder les choses en face, et assurer une plus grande convergence européenne des conditions d'accueil des étrangers. Ce sera notre sixième axe. Nous voulons que la France ne soit ni moins accueillante ni moins attractive que ses voisins. Cela concerne notamment l'accès au système de santé : l'aide médicale de l'État, ou encore les conditions d'accès des demandeurs d'asile à la protection maladie. Des pistes sont à l'étude : la secrétaire d'État Christelle Dubos y reviendra sans doute. Nous aurons sur ce sujet une discussion précise lors de l'examen du projet de loi de finances. Maîtriser les flux migratoires, c'est bien évidemment aussi renforcer notre efficacité dans l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. J'ai parlé de l'action diplomatique. Mais nous avons aussi renforcé nos outils juridiques, avec la loi du 10 septembre 2018. Les éloignements contraints ont ainsi augmenté de 20 % en deux ans. Cette augmentation se poursuit d'ailleurs sur la même tendance en 2019. Mais nous voulons faire mieux, en tirant le meilleur parti des outils que nous nous sommes donnés et en menant un nouvel effort capacitaire, par exemple sur le nombre de places de rétention administrative.

Nous avons créé un outil technique d'appui à l'évaluation de la minorité, pour distinguer les vrais mineurs des demandeurs en réalité adultes, pour lutter contre les fraudes et les détournements. Et nous avons renforcé notre solidarité financière à l'égard des départements en la matière. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin, pour nous assurer que le nouvel outil technique déploie sa pleine efficacité et inciter à son utilisation partout sur le territoire, mais aussi pour redéfinir les critères selon lesquels s'opère à l'échelon national la répartition entre départements des mineurs à accueillir. Nous présenterons des solutions dans les prochaines semaines, dans le prolongement de nos échanges les plus récents avec l'Assemblée des départements de France. J'attire aussi votre attention sur la nécessité d'affiner la réponse qu'il convient d'apporter à certains territoires, notamment les outre-mer. Le Gouvernement n'a pas hésité à décider d'adaptations nécessaires pour répondre à leur spécificité. Ainsi, pour Mayotte, nous avons engagé une action globale de lutte contre l'immigration clandestine qui mobilise les forces armées aux côtés de la police et de la gendarmerie. Cette action globale passe également par une coopération renforcée avec l'Union des Comores. Je veux aussi relever que nous avons décidé d'adapter les modalités d'accès à la nationalité française pour les ressortissants étrangers nés à Mayotte : je salue ici le travail législatif mené au Sénat sur l'initiative du vice-président Thani Mohamed Soilihi. Dans l'océan Indien, nous avons conduit une action de coopération avec les autorités du Sri Lanka pour éviter les départs de migrants depuis ce pays en direction de La Réunion. Je n'oublie pas non plus la Guyane, qui est exposée à un flux important de demandeurs d'asile, dont un très grand nombre sont déboutés. Nous y avons lancé l'expérimentation de la prise de décision en deux mois : le signal a été clair, et les demandes d'asile ont sensiblement diminué. Nous allons étendre ce dispositif aux départements français des Antilles. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne sais pas si les échanges seront aussi vifs ici qu'à l'Assemblée nationale au cours du débat sur l'immigration. Si tel est le cas, j'espère que cette vivacité sera féconde en solutions. Je suis sûr que la Haute Assemblée a une contribution originale à apporter à ce débat, notamment en exprimant le ressenti des territoires et en se faisant l'écho du point de vue des élus locaux. Nos concitoyens ont les yeux rivés sur les réponses que nous apporterons ensemble. L'équilibre et l'efficacité de notre politique dépendront en partie de la qualité des échanges que nous pourrons avoir.

messieurs les sénateurs, j'aimerais partager avec vous quelques convictions sur la politique d'immigration. La première est que notre politique migratoire est, et doit être une question globale.

Parler d'immigration, c'est souvent parler aussi de sa propre histoire, avec son propre vécu. Parler d'immigration, c'est évoquer un sujet qui touche chacune et chacun d'entre nous. Nous devons l'aborder par les faits, en nous tenant éloignés des et des idées reçues, qui sont Notre politique d'immigration, c'est d'abord une question internationale. Et c'est au coeur de cet ordre international que se trouve un acteur absolument incontournable sur la question migratoire : l'Europe. D'abord, c'est la question de Schengen. Schengen, vous le savez, s'est construit sur deux piliers : la libre circulation des personnes à l'intérieur des frontières et la protection des frontières extérieures. Malgré des avancées fortes, indéniables, puissantes sur le premier pilier, jusqu'à il y a peu, le second n'avait été qu'insuffisamment traité. Malgré des contrôles extrêmement stricts dans certains points, quelques frontières extérieures de l'Union européenne, que nous appelons des « frontières vertes », sont encore insuffisamment contrôlées. C'est pour cette raison que le Président de la République s'est engagé très tôt pour la réforme de Schengen, notamment afin d'encourager l'établissement de centres contrôlés aux frontières extérieures de l'Europe, de mieux nous appuyer sur l'Agence européenne de garde-frontières et de créer une Agence européenne de l'asile, enfin, de poser la question de la prise en charge financière des procédures. Corolaire nécessaire de cette réforme de Schengen, nous devons revoir nos règles en matière de droit d'asile. Fixant un principe en apparence simple- le pays de première entrée d'un demandeur d'asile traite sa demande -, le règlement Dublin s'est révélé

Si on ajoute à cela les demandes multiples introduites par les demandeurs d'asile et l'action innommable des trafiquants d'êtres humains, les principes de solidarité entre les États membres ont été totalement compromis. Pourtant, il est possible de les faire vivre. J'étais la semaine dernière à La Valette avec plusieurs de mes homologues européens. Nous avions des intérêts parfois divergents, mais nous avons trouvé des premières solutions ensemble. Au conseil des ministres « justice et affaires intérieures » d'hier, où Amélie de Montchalin représentait la France, nous avons exposé notre souhait de poursuivre cette dynamique pour mener une réforme globale et durable du système d'asile sur les deux fondements qu'a rappelés le Premier ministre : solidarité et responsabilité. En effet, dès l'installation de la nouvelle Commission européenne, nous devons être prêts à proposer des solutions pour avancer sur la refondation de Schengen et sur la réforme du régime d'asile européen. Mesdames, messieurs les sénateurs, la France sera au rendez-vous. La responsabilité, cela signifie que des règles effectives doivent déterminer les compétences respectives des États membres pour l'examen des demandes d'asile. Certains pays ont plaidé pour une augmentation de la durée de responsabilité. Celle-ci devra naturellement s'effectuer dans une proportion raisonnable. Pour réduire les mouvements secondaires, nous rechercherons des solutions en proposant par exemple qu'un demandeur d'asile ne puisse bénéficier des conditions matérielles d'accueil que dans un seul État, est responsable de sa demande. La solidarité, cela signifie qu'une gestion ordonnée des migrations à l'échelle de l'Europe suppose que nous cherchions à aider vraiment les États de première entrée. La France se prononcera en faveur d'un mécanisme de solidarité, solidarité, qui devra être obligatoire. Obligatoire dans son principe, cette solidarité pourra bien entendu se manifester par des formes différentes selon les États. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous ne pouvons pas envisager notre politique d'immigration sans connaître ce contexte européen, mais nous ne pouvons pas débattre sans partir des faits. Le premier fait que je veux évoquer, ce sont les Le premier fait que je veux évoquer, ce sont les entrées régulières sur notre territoire. En 2018, 256 000 personnes sont arrivées régulièrement. Parmi elles, 90 000 sont arrivées par la voie de l'immigration familiale ; ce chiffre est stable depuis de longues années.

256 000, c'est deux fois plus que la demande d'asile, sur laquelle, bien souvent, nous nous arrêtons. Mais il faut noter que la demande d'asile en France présente plusieurs singularités. La première, c'est son augmentation. Il y a eu, l'année dernière, 123 000 demandes d'asile en France : c'est un record, et cela représente une hausse de 20 % par rapport à 2017, alors même que la demande d'asile en Europe a significativement baissé. fortement dans certains pays : en Allemagne, la baisse est de 18 % sur la même période. Ces données doivent nous conduire à nous interroger, car elles ont des conséquences sur nos capacités à instruire convenablement les demandes et à traiter dignement celles et ceux qui ont besoin de protection.

Elle recense les pays où l'État de droit est garanti, où l'État n'est pas une menace pour ses citoyens. Ainsi, aujourd'hui, un quart de notre demande d'asile provient de pays dits « sûrs », notamment de Géorgie et d'Albanie, deux pays depuis lesquels la demande est en forte augmentation. À ces demandes s'ajoute la défaillance du système Dublin, puisque 30 % des demandes d'asile effectuées le sont par des personnes ayant déjà introduit une demande dans un autre pays Ces chiffres ont donc un sens, que nous devons affronter : il est possible que notre système d'asile soit en partie dévoyé, détourné. Et l'on constate qu'une pression très forte s'exerce sur nos services publics, notamment les préfectures ou notre système de santé. Nous avons pris les choses en main, singulièrement en augmentant nos capacités d'hébergement pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Nous nous sommes aussi emparés, dès le début du mandat, des questions d'immigration, d'asile et d'intégration. La loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a été une première étape. Elle est aujourd'hui pleinement entrée en vigueur. Toutes les mesures réglementaires nécessaires à son application ont été prises et les crédits budgétaires, les moyens matériels, humains et les mesures d'organisation ont été au rendez-vous. Ce texte a permis des avancées fortes, nécessaires, utiles. Je pense notamment à l'allongement de la durée maximale de rétention de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours, qui a permis des éloignements que nous n'aurions pas pu réaliser autrement. Je pense également à la possibilité offerte aux préfets de prendre dans certains cas des mesures d'éloignement après une décision de l'Ofpra confirmée par les juridictions. Depuis son entrée en vigueur, 3 000 OQTF- obligations de quitter

Je veux dire aussi que Laurent Nunez et moi-même multiplions les déplacements pour améliorer nos coopérations avec les pays d'origine. Nous utilisons également toutes les options qui nous sont offertes pour lutter contre l'immigration irrégulière,

Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux le dire fermement : nous pensons notre politique d'immigration pour réussir notre politique d'intégration. Sur ce point, notre gouvernement s'est engagé fortement. Les crédits budgétaires dévolus à l'intégration ont été portés à des niveaux sans précédent

Nous avons renforcé les programmes qui favorisent l'insertion professionnelle. Ils font désormais pleinement partie de nos politiques d'intégration et nous devons aller plus loin encore, notamment pour les femmes ou les réfugiés qualifiés. À cette fin, nous avons engagé une réflexion pour simplifier les procédures et revoir la liste des métiers dits « en tension ». Enfin, nous devons prendre en compte le désir exprimé par de nombreux réfugiés de résider dans les grands centres urbains. C'est une difficulté de gestion supplémentaire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la question de notre politique migratoire est une clé pour notre pacte républicain, une clé pour notre intégration, une clé pour la confiance entre les dirigeants et les Français. Nous ne transigerons pas sur nos valeurs. Nous aborderons toutes les solutions avec sérieux et sérénité, sans caricature. Le Premier ministre a dessiné quelques pistes lundi à l'Assemblée nationale ; elles se précisent Nous avons besoin de regarder cette question en face, sans passions excessives ou fantasmes entretenus. Nous avons besoin de faire preuve de courage, d'avancer des propositions et d'aborder tous les aspects du débat, sans exception. La parole

le Gouvernement a tenu à ce que ce débat sur les politiques migratoires puisse avoir lieu devant la représentation nationale, d'abord, et avant tout, parce que cette question est un sujet de préoccupation pour nombre de nos concitoyens et élus que vous

Je concentrerai mon propos sur sa perspective internationale, en particulier européenne. Nous avons, tout d'abord, besoin de clarté sur la situation réelle des migrations vers l'Europe et vers la France. Les mouvements migratoires vers l'Europe diminuent. Ainsi, alors que le nombre d'entrées irrégulières sur le territoire de l'Union européenne s'élevait à 1 820 000 en 2015, il est retombé à 180 000, soit dix fois moins, en 2018. Et pour 2019, la baisse est actuellement de 29 % par rapport à l'an dernier. Pour autant, le sujet reste d'actualité : en Europe, nous le savons, les flux peuvent reprendre, car la situation géopolitique n'est pas stabilisée en Syrie. Je saisis d'ailleurs l'occasion pour condamner très fermement l'offensive turque au nord de la Syrie.

est mis à l'épreuve. Il nous faut agir, maintenant. Agir pour conserver notre capacité à accueillir dans les meilleures conditions ceux qui ont droit à l'asile dans notre pays ; agir pour pouvoir continuer à intégrer à notre société ceux qui viennent d'obtenir la nationalité française ou un titre de séjour régulier ; surtout, agir en Europe. Si nous n'agissons pas, nous risquons de voir l'espace Schengen imploser et l'Europe se défaire. Les Européens doivent avancer ensemble sur ce sujet sans attendre qu'une nouvelle crise se profile. Il ne peut y avoir parmi les États membres européens certains qui choisissent la résignation, d'autres qui choisissent l'indifférence. Nous devons être capables de nous organiser pour faire preuve d'humanité à l'égard de ceux qui demandent protection et d'une absolue fermeté contre les trafiquants et les passeurs qui exploitent la détresse de ceux qui souffrent.

Notre approche doit prendre en compte l'ensemble des géographies concernées : les pays d'origine et de transit, la Méditerranée et l'Union européenne. Sur ces trois volets, l'Europe a un rôle essentiel à jouer

L'aide publique au développement a bien sûr un objectif propre : la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Mais elle est aussi un levier essentiel de notre politique migratoire, et ce pour trois raisons.

Ensuite, notre aide publique au développement permet à nos partenaires du Sud de se doter des capacités indispensables pour maîtriser eux-mêmes les flux migratoires. On le sait, en effet, le défi migratoire est d'abord un défi pour les pays du Sud, et tout le sens de notre action est de les aider à y faire face. Enfin, l'aide publique au développement est essentielle pour traiter dans la durée les causes profondes des migrations irrégulières. Nous devons aider les populations tentées par l'émigration par désespoir à retrouver des perspectives, un avenir et des conditions économiques de développement, là où elles vivent.

que 10 % de l'enveloppe de ce nouvel instrument de coopération et de développement international soient alloués à ces questions. C'est une priorité des négociations que je soutiens avec mes homologues sur ce budget.

C'est inacceptable ! Nous devons nous mobiliser et, comme l'a rappelé Christophe Castaner, mettre en place un mécanisme de sauvetage et de débarquement efficace Le Président de la République l'a proposé, afin de trouver une solution européenne collective de responsabilité et de solidarité. Des avancées ont été obtenues le 23 septembre à La Valette. Mais les migrations ne sont pas seulement l'affaire de quatre pays, l'Allemagne, l'Italie, Malte et la France.

par certains. Nous devons enfin agir ensemble sur le sol européen. Nous devons poursuivre nos efforts pour mieux contrôler nos frontières extérieures. L'agence Frontex pourra mobiliser 10 000 garde-côtes et garde-frontières dans les prochaines années, afin d'aider les États membres en matière de contrôles frontaliers et de reconduites. Il y a là un enjeu évident de souveraineté européenne. Il faut bien entendu refonder Schengen, qui repose sur deux jambes : la liberté intérieure de circulation et de réels contrôles aux frontières extérieures. Depuis maintenant trente ans, ce système est boiteux : la jambe « liberté intérieure » est forte, mais la jambe « protection de nos frontières extérieures » est faible. Il nous faut donc revoir ce système pour préserver notre liberté de circulation en Europe.

C'est l'un des enjeux de la révision du régime d'asile européen, le fameux règlement de Dublin, qui doit nous permettre d'harmoniser nos systèmes nationaux et de limiter les demandes multiples et parallèles d'asile successivement dans plusieurs pays, qui créent des mouvements secondaires extrêmement difficiles à contrôler. sera l'essentiel de notre action pour les prochains mois. Ursula von der Leyen a annoncé vouloir un pacte sur l'asile et l'immigration. La France est à ses côtés, et je peux vous dire qu'il y a eu aujourd'hui une unanimité en Europe sur le besoin de refonder profondément ces deux piliers : asile et immigration, et espace Schengen. notre modèle d'accueil et d'intégration est, je le crois, l'honneur de notre République. Notre devoir est bien de tout faire pour en préserver la viabilité. En plus d'y consacrer nos politiques nationales, nous y employons, vous le voyez, nos leviers d'action internationaux et européens. Mais pour mieux répondre aux défis migratoires d'aujourd'hui et de demain, nous avons également besoin de vous, élus de nos territoires, et je sais à cet égard la qualité des travaux du Sénat, informés et sérieux, sur les thèmes de nos débats. Je suis donc particulièrement heureuse d'échanger avec vous sur ces sujets, dans la transparence et la responsabilité, sous le regard des Français. La parole

C'est, me semble-t-il, une bonne occasion de tordre le cou à beaucoup d'idées reçues, tout en nous montrant vigilants et fermes quand les situations l'exigent. Si je pense qu'il est important que nous puissions débattre ensemble de cette question, c'est évidemment parce qu'elle interpelle nos concitoyens, mais c'est aussi parce que, pendant plus de vingt ans, comme travailleuse sociale, j'ai été confrontée à tout ce que l'incompréhension et la confusion peuvent provoquer comme rejet de l'autre et comme dégâts pour notre cohésion sociale. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut ouvrir ce sujet à tous nos à tous nos concitoyens, et ne pas le laisser à une seule famille politique qui dupe nos concitoyens avec un discours aussi brutal que simpliste. Dans la foulée d'un grand débat historique, le Président de la République n'a pas éludé la question migratoire, allant jusqu'à affirmer que « le deuxième grand combat européen avec le climat, c'est le combat en matière de migration ». Oui, l'enjeu des migrations dépasse largement les frontières de la France, et l'Europe doit construire cet espace commun, parce qu'une Europe qui sait maîtriser les flux migratoires, ce sont des États membres qui accueillent mieux. Mieux accueillir, c'est respecter des conventions auxquelles la France est partie et dont l'accès aux droits fondamentaux est un pilier essentiel. En France, et nous pouvons en être fiers, chacun, quelle que soit sa situation, peut accéder aux soins. C'est tout le sens d'une protection maladie qui est universelle, puisqu'elle permet à chaque personne qui travaille ou qui réside en France de manière stable et régulière de bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé. En France, votre couverture maladie ne dépend pas de votre emploi ou de votre statut. Cette protection est donc accessible quelle que soit la nationalité de l'assuré, et elle inclut les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour, les réfugiés, mais aussi les demandeurs d'asile. Des dispositifs sont aussi prévus pour la prise en charge des soins des personnes migrantes en situation irrégulière. C'est le cas de l'aide médicale de l'État, l'AME, qui permet de couvrir les soins essentiels des ressortissants étrangers en situation irrégulière, en médecine de ville comme à l'hôpital. Cette couverture n'est pas immédiate, puisqu'elle nécessite une présence d'au moins trois mois sur le territoire. Par ailleurs, elle est délivrée sous condition de ressources. Si ces conditions ne sont pas remplies, la prise en charge est alors limitée à celle des soins urgents. Ces procédures sont indispensables. Agnès Buzyn l'a bien rappelé lundi à l'Assemblée nationale : « en France, on ne laisse pas des personnes périr parce qu'il leur manque le bon tampon sur le bon document. Elles sont aussi indispensables pour des raisons de santé publique et pour éviter la propagation de maladies. L'aide médicale de l'État répond également à un impératif d'économies si elle n'existait pas, elle aurait pour conséquence une dépense plus grande, parce qu'une prise en charge tardive d'une maladie est toujours plus coûteuse qu'une prise en charge à temps par la médecine de ville. Pourtant, certaines caricatures ont la vie dure, et l'aide médicale de l'État n'y échappe pas. Elle est même devenue, au fil des années, un motif récurrent des discours de peur et de repli. Il est temps de clarifier les choses ! Avec l'AME, le niveau de prise en charge est moins important que celui des assurés en situation régulière qui, à ressources égales, bénéficient de la CMU-C. la CMU-C. Ainsi, les actes de PMA, les médicaments à service médical rendu faible, remboursés à 15 %, et, bien sûr, les frais de cures thermales ne sont pas pris en charge par l'AME. Les frais pris en charge en grande partie par les complémentaires santé, tels que les frais dentaires ou optiques, le sont pas par l'AME. Enfin, les soins à visée esthétique ne sont, bien évidemment, pas pris en charge par l'AME. S'agissant des autres droits sociaux, l'objectif est de faciliter l'intégration des personnes. Sur ce sujet, je veux mettre fin, là encore, aux idées reçues, qui voudraient que les étrangers en situation irrégulière aient un large accès aux prestations sociales. Les personnes en situation irrégulière n'ont droit à aucune prestation en dehors de la prise en charge de leurs soins. Je n'inclus pas dans ce propos les demandeurs d'asile, qui ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière sur notre territoire. S'agissant des personnes en situation régulière, nous appliquons des principes constitutionnels et des règles internationales qui s'imposent à tous et par lesquelles se matérialise l'accès aux droits fondamentaux. Ces principes, nous y tenons. Pour autant, l'égalité de traitement n'est pas totale : la plupart des minima sociaux sont soumis à des conditions de résidence plus restrictives pour les ressortissants étrangers en situation régulière que pour les ressortissants français. Par exemple, pour percevoir le RSA, une condition de cinq ans de résidence sur le territoire est requise. Cette différence de traitement n'est pas contraire n'est pas contraire à notre exigence de cibler les besoins des populations concernées, parce qu'il en va de leur santé et de leur intégration. Il ne faut pas oublier que les personnes migrantes sont souvent plus vulnérables : il est donc indispensable d'aller vers elles pour qu'elles puissent accéder aux soins et aux droits. C'est la raison pour laquelle nous avons structuré un parcours de santé des primo-arrivants, en lien avec le secteur associatif, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les agences régionales de santé, pour organiser une prise en charge des besoins le plus rapidement possible. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons augmenté les moyens alloués aux permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, qui réunissent soignants et travailleurs sociaux, accueillent de manière inconditionnelle et exercent cette mission d'accompagnement médico-social des personnes les plus vulnérables. Je profite de ce débat pour saluer le travail remarquable des travailleurs sociaux et des associations, qui oeuvrent chaque jour avec une énergie remarquable au service de cette intégration. Quand certains cultivent une rente en alimentant le rejet, d'autres sont sur le terrain et trouvent des solutions pour que la cohésion sociale soit autre chose qu'une belle expression dans un discours. Pour autant, nous sommes vigilants : comme pour toutes les politiques publiques, nous nous interrogeons sur l'efficience du système et nous ne fermons pas la porte à l'identification d'éventuels abus. Cette démarche est indispensable pour restaurer la confiance dans notre système, qui semble aujourd'hui faire défaut. Je pense en particulier à l'aide médicale de l'État, qui représente une dépense de 848 millions d'euros en 2018. C'est une dépense importante. Pourtant, je rappelle que la dépense par bénéficiaire de l'AME est équivalente à la dépense par bénéficiaire d'un assuré, alors même que l'état de santé des bénéficiaires de l'AME est notoirement plus dégradé. Une mission a donc été confiée aux inspections générales pour faire la lumière sur d'éventuels fraudes ou abus et pour proposer des pistes de progression. Ces pistes pourront tenir compte des modèles en vigueur chez nos principaux voisins, même si, au-delà des comparaisons, c'est bien le cadre de prise en charge le plus pertinent et le plus efficace Plusieurs options sont actuellement étudiées par la mission d'inspection. Nous regarderons l'ensemble des options proposées avec une grande attention, mais je souhaite préciser dès aujourd'hui que nous ne retiendrons pas la solution d'une participation financière des personnes admises à l'AME cela constituerait un obstacle trop important pour l'accès effectif aux soins. L'introduction éphémère d'un droit de timbre en 2011 a montré qu'une telle mesure ne faisait que reporter les coûts de prise en charge sur les soins urgents. Deux autres pistes sont étudiées par la mission d'inspection : subordonner à un accord préalable l'accès à certaines prestations, en dehors des soins urgents ou vitaux ; ajuster le périmètre du panier de soins pris en charge par l'AME. Mais encore une fois, ce ne sont que des pistes, et nous attendons que la mission rende ses conclusions à la fin de ce mois. En revanche, nous n'attendons pas les conclusions de cette mission pour renforcer les contrôles : l'AME et les soins urgents ne doivent pas être détournés de leur vocation, et ils doivent bénéficier à ceux qui y ont effectivement droit. Ces contrôles portent sur les conditions d'éligibilité à l'AME, comme la durée du séjour et les ressources effectives des demandeurs, mais peuvent également avoir lieu, en particulier pour ce qui concerne les bénéficiaires qui ont le plus recours aux soins. Le regroupement des demandes d'AME dans trois caisses primaires d'assurance maladie permettra de mieux les contrôler. Nous allons ainsi déployer un plan de lutte contre les fraudes. L'une des mesures de ce plan permettra de lutter contre le phénomène des détournements de procédure de ressortissants étrangers bénéficiant d'une assurance privée dans le cadre d'un visa Schengen, mais qui demandent l'AME pour bénéficier de soins considérés comme étant de meilleure qualité Les caisses d'assurance maladie auront accès, dès la fin de l'année, à la base Visabio du ministère de l'intérieur, qui permettra d'identifier les demandeurs dissimulant un visa et n'ayant donc aucunement vocation à bénéficier de l'AME ou des soins urgents. Voilà de manière très concrète et pragmatique comment nous voulons redonner confiance dans un système auquel nous sommes très attachés. S'agissant du cas particulier des demandeurs d'asile, le régime est celui d'une affiliation à l'assurance maladie, et donc souvent à la CMU-C, dès le dépôt de la demande. Une hausse significative de demandes d'asile a été observée par des personnes en provenance de pays signalés « d'origine sûre », ce qui signifie que dans l'immense majorité des cas, ces demandes d'asile n'aboutiront pas. L'abus est par conséquent rendu possible par cette affiliation immédiate à l'assurance maladie. Seule une étude approfondie nous permettra d'en savoir plus sur l'existence de ces filières et donc de repenser, si cela est nécessaire, les conditions d'affiliation à l'assurance maladie pour les demandeurs d'asile. Cette étude est en cours et la mission d'inspection est au travail. Un délai de carence, pendant lequel nous prendrions évidemment en charge les soins urgents, pourrait se concevoir, comme c'est le cas d'ailleurs pour les Français qui rentrent de l'étranger sans activité professionnelle. Lutter contre les fraudes, c'est mettre fin à une suspicion qui nuit à tous les autres : ce n'est pas remettre en question notre obligation constitutionnelle d'un accès à la santé pour tous. C'est surtout le moyen le plus sûr de mettre enfin un terme aux idées fausses qui circulent. Mesdames, messieurs les sénateurs, faire vivre les grands principes sans être naïfs, c'est être fidèles à nos valeurs sans laisser prospérer des discours de peur. Notre exigence doit être celle de la justice envers les populations vulnérables, pour que la manière dont nous les accueillons soit conforme à l'image que nous nous faisons de la grandeur de la France. Dans la suite

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, mesdames les secrétaires d'État, mes chers collègues, le Président de la République, devant les parlementaires de la majorité, s'est livré à une action de populisme d'État qui a étonné et choqué.

de procédures ! Toutes les migrations sont légitimes, mes chers collègues. Mais l'asile, qui protège le combattant de la liberté, la personne menacée dans son existence, est un droit, un engagement et un devoir pour notre nation. Nos principes constitutionnels et nos engagements conventionnels sont une partie de nous-mêmes. Ainsi, toutes les migrations ne peuvent pas être mises sur le même plan. Pour déterminer si une personne relève de la convention de Genève, une instruction de sa demande doit être diligentée. L'asile est un droit quand l'immigration est une politique- il faut bien séparer les choses. Mais l'immigration est aussi une richesse. Elle a accompagné notre pays dans ses années de croissance. D'ailleurs, le Canada, qui n'a pas oublié qu'elle était une richesse, continue à prospérer

ou alors le droit du sol avec action volontaire, avec conditions de scolarité et de stage. C'est très différent ! Il ne faut pas laisser croire aux gens qu'il suffit de naître en France pour devenir français ... De la sorte, on se retrouve avec la situation de Mayotte

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le président,

La question migratoire nourrit de nombreux populismes, en France, comme chez certains de nos voisins. Elle entraîne même de dangereuses fractures au sein de l'Union européenne. Pour notre part, nous abordons ce débat en toute responsabilité, sans angélisme ni aveuglement, forts des valeurs de dignité que nous avons toujours défendues. Cette question est effectivement complexe ; elle confronte nos sociétés à des défis, inédits dans leur ampleur comme dans leur durée. Depuis le pic migratoire de 2015, le nombre d'arrivées aux frontières de l'Europe a fortement faibli, cela a été rappelé. Hélas, ce reflux n'évite pas de nouvelles tragédies comme, encore récemment, la noyade de dix-huit personnes au large de Casablanca. Nul ne peut évidemment rester insensible face à de tels drames, ce qui ne doit pas nous interdire d'aborder aussi la question migratoire sous l'angle de la sécurité, de la politique intérieure et de l'intégration. Pour autant, le premier facteur des migrations est économique ou, pour le dire autrement, lié au besoin fondamental de vivre dignement. Ainsi, bien que le taux d'extrême pauvreté dans le monde ait été divisé par quatre depuis trente ans, 800 millions de personnes vivent encore dans un dénuement total. On compte encore trop d'États faillis ou en proie à des conflits de haute intensité pour envisager un tarissement des flux de réfugiés. N'oublions pas non plus que les migrations climatiques ne feront qu'augmenter. Dans ces conditions, il est évident que pour nombre de ces femmes et ces hommes, migrer est avant tout une nécessité vitale.

est, semble-t-il, en préparation. La politique migratoire comporte deux axes : la lutte contre l'immigration irrégulière, en lien avec les pays de départ, et la politique d'accueil et d'intégration sur notre sol. Le premier axe, qui se déploie à l'échelle européenne, a porté ses fruits en réduisant, je l'ai dit, les flux. Depuis 2015, l'Union européenne a mis en oeuvre un certain nombre de mesures, que mon groupe a approuvées pour la plupart accord avec la Turquie en mars 2016, mise en place des hotspots, création du centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants et, bien sûr, les dispositifs de relocalisation. Néanmoins, le Conseil européen avait préconisé, à la fin de l'année 2018, d'accentuer la lutte contre les trafiquants. Où en est-on sur ce point ? Qu'en est-il du renforcement du mandat de l'agence européenne ayant remplacé l'agence Frontex, en particulier du déploiement des garde-frontières et des experts en matière de retour ? S'agissant de l'accueil des migrants, certains points font certes polémique, mais, derrière, se trouvent des questions légitimes. Sommes-nous capables d'offrir un accueil digne aux personnes arrivant en France ? Comment bien accueillir, en fonction de nos capacités, pour permettre une réelle intégration ? À notre sens, rien ne doit être tabou : tout dispositif peut être discuté tant qu'il s'inscrit dans les valeurs et principes de notre République. Je pense, en particulier, à l'aide médicale de l'État, à laquelle l'ensemble de mon groupe reste profondément attaché. D'abord, elle participe du droit inaliénable à la santé pour toute personne. Ensuite, elle contribue à la protection des populations en tant qu'instrument de prévention des maladies contagieuses. Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. sommes pas naïfs. Notre générosité n'est pas illimitée et nous ne pouvons balayer d'un revers de main l'idée de réformer ce dispositif, pour mieux le calibrer et lutter contre les abus. Pour notre part, nous attendons les conclusions de la mission d'inspection mandatée par Mme la ministre des solidarités et de la santé. Le regroupement familial est, lui aussi, souvent pointé du doigt, pour de mauvaises raisons. Les chiffres sont en réalité très stables depuis 2013, au moins- on observe même une légère baisse -, et se situent autour de 90 000 admissions par an, sur un total de 256 000 titres de séjour délivrés en 2018. Durcir d'un coup les conditions du regroupement familial n'est certainement pas la bonne solution pour réguler l'immigration légale, d'autant que nous sommes également liés par des engagements bilatéraux et internationaux. Sommes-nous condamnés à ne rien faire ? Je ne le crois pas. Peut-être pourrions-nous explorer des pistes d'évolution respectueuses de nos principes, par exemple en introduisant, comme en Allemagne, le critère d'une maîtrise minimale de la langue française ou en renforçant le contrôle du respect par le candidat au regroupement familial des valeurs de la République.

S'agissant du droit d'asile, il est certain que des marges d'amélioration existent quand on sait qu'une partie des demandeurs vient de pays sûrs. Le cas des ressortissants albanais et géorgiens est souvent cité. On peut en tout cas se féliciter de l'amélioration du traitement des dossiers, ainsi que de l'augmentation des capacités d'hébergement des demandeurs d'asile, même si nous devons mieux faire. Néanmoins, aucune réponse ne sera pérenne si elle ne s'inscrit pas dans un cadre européen. Le règlement de Dublin qui permet de se défausser sur quelques pays en première ligne, notamment l'Italie et Malte, n'est pas digne de la solidarité européenne, malgré les petits arrangements consentis au fil de la crise migratoire. Mes collègues du RDSE et moi-même espérons que l'accord de répartition qui s'est dessiné à la fin du mois de septembre à La Valette, distinguant les demandeurs d'asile des réfugiés économiques, aboutira concrètement. Enfin, mes chers collègues, je m'exprimerai en tant que corapporteur, avec Yvon Collin, du budget de l'aide publique au développement. Aider les pays d'origine des migrants est une nécessité à deux égards d'établir des coopérations pour la gestion des frontières des pays de départ, mais aussi de renforcer les soutiens apportés au développement des pays offrant peu d'espoirs à leurs concitoyens. Les priorités se situent essentiellement en Afrique subsaharienne, ce dont nous rediscuterons dans le cadre du très attendu projet de loi d'orientation et de programmation de l'aide au développement. S'agissant du niveau de l'aide, avec nos 0,44 % du revenu national brut, nous sommes encore loin de l'objectif de 0,7 % défini par le Comité d'aide au développement de

Mes chers collègues, dans un monde de plus en plus ouvert, les migrations ne cesseront jamais. Notre pays s'enorgueillit de sa tradition d'accueil, conforme à ses principes humanistes. Toutefois,

ni angélisme ni catastrophisme, mais plutôt un humanisme réaliste

est, je crois, nécessaire pour clarifier nos choix collectifs. Tenons-le à la bonne hauteur et faisons-en un guide partagé de notre politique

Une limitation et une régulation des entrées sont de la nature même des missions d'un État souverain. Tous les pays neufs dans l'histoire qui se sont peuplés par l'immigration, sur le modèle des États-Unis dès le XVIII siècle, ont fixé des limites au droit d'entrée, en les adaptant suivant les périodes et suivant la consolidation de leur société. Nous-mêmes, aujourd'hui, avons tous conscience de la nécessité de faire respecter de telles limites à l'accès à notre sol, pour maintenir les équilibres humains et la cohésion de notre société. Seules des doctrines extrémistes réclament l'abolition de toute frontière et tout contrôle territorial, étant observé, d'ailleurs, que ceux qui les défendent ne sont pas parmi les plus pacifiques lorsqu'ils défilent dans nos rues. Cette régulation est la condition pour que la France assure avec succès l'intégration républicaine, qui est notre tradition et reste notre impératif pour garantir à nos compatriotes une société ouverte et solidaire. L'immigration sous ses diverses formes représente entre 250 000 et 320 000 personnes par an, suivant l'estimation que l'on peut faire des entrées irrégulières. C'est le même ordre de grandeur

Notre connaissance, à tous ici, des réalités locales nous fait bien percevoir que ce chiffre de nouveaux arrivants est un facteur de tension dans le secteur du logement- tout particulièrement à la périphérie des grandes villes -et pèse sur nos principaux services publics, à commencer par l'enseignement et la santé. La régulation du nombre d'entrants est donc une condition première d'une intégration accomplie pour chaque personne admise sur notre sol. Nous pouvons constater une large convergence sur ce principe simple. Les divergences apparaissent, d'abord quand on cherche à estimer le nombre préférable, et surtout quand on veut décider et appliquer les moyens concrets qui seront employés pour écarter les entrées dont nous ne voulons pas et que nous devons refuser. À ce sujet, je souhaite marquer une distance, monsieur le Premier ministre, face à l'idée de quotas d'immigration qui revient encore. La plus grande part des entrées sur notre sol est issue de processus de rapprochement familial, d'accès aux études supérieures et d'asile politique.

Les points noirs de notre situation se situent à trois niveaux : le traitement des demandes d'asile, le mouvement des mineurs isolés et la coordination européenne insuffisante dans l'espace de libre circulation. L'asile politique est une obligation souscrite par notre pays, comme par 140 autres, pour protéger les personnes menacées dans leur vie par la violence régnant dans leur pays. Nous ne pouvons faillir à cette obligation, qui répond impérativement à nos engagements et aux fondements humanistes de la République. En revanche, la lucidité élémentaire nous oblige à constater que chaque année les deux tiers des demandes d'asile présentées en France se révèlent injustifiés après, pourtant, un examen scrupuleux par l'Ofpra et par la justice, avec d'extrêmes garanties de droits de la défense. Or ce n'est pas un hasard malencontreux. La plupart de ces demandes injustifiées sont présentées pour obtenir en réalité une voie d'immigration non contrôlée. L'abus organisé du droit d'asile est un défi à notre système de droit, auquel nous avons le devoir de remédier, faute de quoi l'exercice de ce droit d'asile sera lui-même atteint. Le déroulement de l'examen des demandes, la situation dans laquelle sont placés les demandeurs pendant la procédure et les modalités de leur contrôle sont à réexaminer encore plus rigoureusement. Car la situation actuelle, certes en évolution, aboutit à ce qu'une grande majorité des personnes dont la demande d'asile est injustifiée et rejetée se maintiennent sur le territoire en toute irrégularité. C'est un effectif compris entre 50 000 et 70 000 personnes, chaque année, qui se trouve installé sur notre territoire sans remplir aucune des conditions requises. Nous ne devons pas laisser se perpétuer un circuit de fraudes, minant l'application de tout notre droit. Nous avons légiféré pour rétablir la norme. Nos voisins de l'Union européenne à un tel phénomène de détournement- en tout cas pas avec la même ampleur. Nous devons donc, avec vous, mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, poursuivre nos efforts pour une véritable application de la loi sur l'asile. sur l'asile. Autre source préoccupante d'entrées irrégulières, le mouvement des mineurs isolés est aussi, de manière massive, le résultat de l'activité de filières organisées. Ce n'est pas par une démarche individuelle et improvisée que des milliers de jeunes détruisent leurs documents d'identité, juste après avoir franchi le contrôle à l'aéroport, et se dirigent directement vers le service d'aide à l'enfance, dont l'adresse est enregistrée sur leur téléphone portable. La manière purement sociale dont nous essayons de gérer cette fraude organisée ne peut suffire.

comme je le crois, quelles méthodes conformes au droit ont-ils mises au point qui nous seraient inaccessibles ? Dans ces deux domaines, il n'est pas viable que nous continuions à énoncer une politique largement partagée et que nous échouions à la concrétiser. J'en termine J'en termine par le sujet, trop large pour notre temps de débat de ce jour, du rapprochement entre Européens. Je voudrais simplement, sans casser l'ambiance, insister sur une réalité contrariante il s'agit d'une compétence souveraine des États de l'Union européenne qui n'a été mise en partage communautaire par aucun traité. Absolument ! Nous pouvons tous, en choisissant des mots rassurants- je les ai encore entendus -, parler de « politique européenne » de telle ou telle composante de l'immigration.

pour faire converger un contrôle digne et équitable de l'immigration avec la libre circulation dont jouissent nos 460 millions de concitoyens. C'est un travail contraignant, lent

fixant des principes clairs d'ouverture et en combattant lucidement les mécanismes qui cherchent à les contourner. Si le débat d'aujourd'hui nous aide à clarifier ces principes, en dialoguant de façon rationnelle et tolérante entre nous et avec l'exécutif, nous aurons accompli notre devoir : éclairer l'avenir du pays

monsieur le ministre, mesdames les secrétaires d'État, mes chers collègues, « l'immigration est une chance pour la France ! » Telle est depuis une trentaine d'années la devise, sinon de la République, du moins d'une classe politique qui a tout renié, jusqu'à laisser mourir l'identité du peuple français. Regroupement familial, effacement des frontières, discrimination positive à l'embauche, assistanat social, ... Ah ! ... droit d'asile, faux mineurs mais vrais clandestins majeurs : vous avez créé toutes les conditions d'une véritable submersion migratoire. Alors, l'immigration est une chance, mais pour qui ? Assurément pas pour nos compatriotes. Pour une caste politique, elle a permis de sauver quelques élections grâce à ces nouveaux Français. Pour d'autres, elle a permis de recevoir des subventions publiques et d'affréter des bateaux pour ramener des clandestins des côtes libyennes jusqu'en Europe. Les chiffres sont éloquents : en 2016, seuls 7 % des étrangers qui se sont installés chez nous étaient munis d'un contrat d'embauche. L'immigration n'est plus, et depuis longtemps, une immigration de travail, mais une immigration de peuplement pour assistés sociaux. Pour nos compatriotes, la facture est exorbitante. Je vous le dis solennellement, mes chers collègues, je ne crois pas à la théorie du grand remplacement. En revanche, je suis convaincu de sa réalité. Je n'évoquerai pas, moi, « le bruit et les odeurs » si chers au Président disparu, mais ces zones qui se comptent par centaines à travers le pays et qui sont devenues des enclaves étrangères, des zones de non-France où la haine de tout ce qui est français se répand comme une traînée de poudre. Nos lois, notre culture, notre identité, notre savoir-vivre, notre savoir-être, nos libertés- celles des femmes en particulier -, comme les libertés sexuelles et religieuses, ... Celles que vous n'avez jamais défendues ! ... sont rejetées, combattues, pour être, elles aussi, remplacées sous les coups d'un communautarisme islamiste militant. L'idéologie du vivre ensemble s'écroule sous le poids de la réalité d'une immigration chaque jour plus violente et conquérante, qui met en danger notre unité nationale et républicaine. Seuls ceux qui en ont les moyens en réchappent, et parmi ceux-là, vous tous ou presque mes chers collègues ! Car si la classe politique est favorable au vivre ensemble, elle ne s'inflige pas le « vivre avec ». L'immigration, c'est comme les éoliennes : ceux qui en défendent l'installation refusent d'en voir à côté de chez eux. votre politique d'immigration a aussi le coût du sang. Du Bataclan à Nice, de Laura et Mauranne à Thimothy ou à Théo, c'est notre jeunesse qui est sacrifiée sur l'autel d'une idéologie destructrice. Sur le plan social, la politique d'immigration relève de la provocation. Alors que chaque jour de nouveaux sacrifices sont exigés des Français, l'immigration continue d'être un tonneau des Danaïdes. Le coût de l'AME, qui bénéficie aux seuls clandestins, est passé de 400 millions d'euros il y a quinze ans à 1 milliard d'euros aujourd'hui. Les Français ne s'y trompent plus, ou plutôt vous ne les trompez plus. Ils sont majoritaires à refuser ce suicide national. Les Français en ont marre, les Français en ont assez ans qu'ils se poussent, qu'ils consentent des sacrifices, qu'ils accueillent « l'autre », et qu'ont-ils obtenu en retour ? Le développement d'un insupportable racisme anti-Français, anti-blancs, anti-chrétiens Nos compatriotes refusent la submersion. Ils refusent de devenir des étrangers dans leur propre pays : alors, vous menacez, vous censurez, et vous traînez devant les tribunaux ces résistants qui refusent de collaborer. Comment pouvez-vous avoir les yeux aussi grand fermés devant ce phénomène unique dans l'histoire de l'humanité et des nations : l'explosion démographique mondiale ! Loin d'en prendre conscience, et fidèle à son « en même temps », Emmanuel Macron parcourt l'Europe pour sanctionner les pays qui refusent les quotas de migrants,

longtemps, et je persisterai, même si cela doit me coûter une mise en examen, comme c'est le cas aujourd'hui : car, dans ce beau pays de France, un parlementaire qui dénonce un trafic d'êtres humains se retrouve devant les tribunaux

Les seules questions qui devraient vous animer sont celles-ci : avons-nous, nous, Français, le droit de vivre en France selon nos traditions et notre identité ? Avons-nous le droit de rester ce que nous sommes et de transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents ? Avons-nous le droit de demeurer français dans une France française ? Nous connaissons la réponse, et le sursaut national ne peut donc venir d'aucun d'entre vous : aussi, pour toutes les victimes de votre folle politique d'immigration, pour les victimes sociales, économiques et identitaires, pour toutes ces familles dont la vie a été détruite sous les coups de l'immigration sauvage, je vous demande, mes chers collègues, de droite comme de gauche, car vous êtes tous responsables de ce désastre, je vous demande de vous excuser ! Mais bien sûr ! Excusez-vous pour avoir menti

Excusez-vous en inversant le courant de l'immigration ! C'est terminé ! Si vous refusez, si vous ne renoncez pas à votre idéologie mortifère, bien avant la postérité, c'est la France qui vous maudira

pas besoin de trouver un justificatif pour ce débat. Alors, on peut s'interroger. Que s'est-il passé depuis le vote de la dernière loi ? Pourquoi proposer un débat sous ce format précis ? Est-ce pour revenir sur les dispositifs les plus graves de la loi Collomb, tels que la suspicion généralisée à l'égard des demandeurs d'asile et la multiplication du recours à l'enfermement administratif, y compris d'enfants, ou encore les expulsions vers des pays en guerre ? Est-ce pour améliorer les conditions d'accueil dans les préfectures ? Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté lundi à l'Assemblée nationale et cette après-midi au Sénat : visiblement, ce n'est pas le cap voulu. En résumé, la dernière loi adoptée en matière d'immigration était déjà très dure, et vous venez aujourd'hui nous expliquer comment être encore plus dur. Je ne m'y attarderai pas longtemps, mais les visées politiciennes et électoralistes évidentes que recèle ce débat sont dangereuses : comme on l'a encore entendu il y a quelques secondes, elles ouvrent les vannes de logorrhées haineuses, violentes, vulgaires, mêlant sans vergogne religion et nationalités, de la part de négationnistes et de personnages condamnés pour propos racistes. Mais revenons à notre sujet. La crise économique, sociale et environnementale que traverse notre pays est profonde. Elle provoque colère et angoisse, à l'origine en particulier du mouvement des « gilets jaunes le fameux grand débat national nous aura au moins enseigné ceci : les questions migratoires sont loin d'être parmi les premières préoccupations des Français ces Français que le Président de la République essaie d'opposer aux immigrés, bien sûr responsables de tous les maux des classes populaires, qui en seraient les victimes, les bourgeois étant exonérés de tout soupçon raciste Au-delà du mépris indécent que révèlent de tels propos, ce discours est pour le moins simpliste, les immigrés constituant aussi le tissu social des classes populaires. S'il voulait se soucier des classes populaires, le Président de la République ferait mieux d'agir pour développer les services publics, pour améliorer d'urgence les conditions de vie, en termes de logement, de santé, de transports par exemple, et pour lutter contre la précarité et le chômage dans nos territoires, notamment en Seine-Saint-Denis. Je

mais, pour moi, ce n'est pas un problème. Pour relancer ce débat, vous agitez et manipulez les chiffres du droit d'asile. François Héran, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire migrations et sociétés, considère pour sa part que, s'il y a problème, c'est parce que le diagnostic initial est faux : la France est loin, très loin d'être le premier pays d'Europe pour la demande d'asile. « Raisonner en chiffres absolus n'a aucun sens quand il s'agit de comparer des pays de taille inégale et de richesse variable. » Ainsi, en passant des chiffres bruts aux chiffres relatifs, les 400 000 demandes enregistrées sur notre sol depuis janvier 2015 ne représentent que 10 % du total européen ; et, dans l'hypothèse où toutes les personnes concernées seraient restées en France, elles n'auraient accru notre population que de 0,6 %, contre 2 % en Allemagne moyenne dans l'Union européenne. Aussi, à l'échelle de l'Europe, vu notre population et notre économie, on se fourvoie quand on imagine que des facteurs d'attraction exceptionnels, comme l'aide médicale de l'État ou le regroupement familial, placeraient notre pays en première ligne.

Après le « shopping de l'asile », La République En Marche et le Gouvernement nous ont parlé de « tourisme médical ». Mais sachez que toute mesure qui contribue à réduire l'accès de toutes et tous à la santé est contraire au respect des droits fondamentaux et porte atteinte à la dignité individuelle. De plus, ces choix soulèvent d'importantes questions en matière de santé publique. La ministre, Mme Agnès Buzyn, se veut rassurante sur le sujet, mais, quand même, ne soyons pas dupes : les conclusions des rapports demandés aux inspections concernées seront la sécurité sociale ... Nous veillerons aux mesures qui seront alors adoptées. Tous ces reculs proposés à l'échelle nationale ne sont bien sûr que le reflet de la politique migratoire européenne en vigueur. L'approche uniquement sécuritaire de l'immigration défendue par l'Union européenne n'est plus à démontrer : elle est parfaitement assumée depuis la création de l'agence Frontex, que vous n'avez de cesse d'encenser, sans parler des accords avec la Turquie, conclus à la suite de la crise syrienne. Dans ce cadre, deux points doivent être soulevés à l'échelon européen. Premièrement, la définition des « pays d'origine sûrs » doit être revue. Je pense évidemment au prétendu détournement du droit d'asile, dont vous parlez en boucle, par les Albanais et les Géorgiens. L'asile n'a été accordé qu'à 8 % des Albanais et à 5 % des Géorgiens pourchassés bien souvent pour des raisons de vendetta, d'orientation sexuelle ou même d'engagement politique, comme le rappellent la Cimade ou bien peu sûrs figurent sur cette liste : je songe par exemple au Bénin. Qu'en pensez-vous ? Deuxièmement, le règlement de Dublin, dont vous appelez de vos voeux le renforcement, est obsolète. Un autre système doit le remplacer. À plusieurs reprises, le Défenseur des droits a appelé le Gouvernement à suspendre l'application de ce règlement pour permettre à des personnes extrêmement fragilisées par des mois d'errance de demander l'asile. Il rappelle qu'il existe, « en Europe, plusieurs centaines de milliers de personnes dont le retour dans le pays d'origine- du fait de leur nationalité -est impossible mais qui, en application de ces règles, ne trouveront jamais d'issue juridique et humaine à leur situation. Or, en 2017, la France s'est révélée la championne européenne des refus d'entrée aux frontières terrestres, renvoyant massivement des personnes en quête de protection vers l'Italie. Quoi qu'il en soit, la question de l'immigration se posera de nouveau très rapidement, et dans des termes internationaux. Il nous faudra alors défendre une interprétation plus large des critères de la convention de Genève, notamment pour tenir compte des nouvelles causes d'exil forcé, qui affectent des groupes entiers de personnes, comme les conséquences du dérèglement climatique. Le fait de renforcer les opérations de police aux frontières et la politique d'expulsion ne changera rien à cet état de fait, pas plus que l'instauration de quotas révélateurs d'une vision néocolonialiste et assez étroite de nos frontières.

les riches vont où ils veulent à tire-d'aile, les plus pauvres vont où ils peuvent en ramant, ceux qui ont la maîtrise des stocks [ ...] peuvent jouer avec les flux en devenant encore plus riches, ceux qui n'ont rien en stock sont les jouets des flux.

pour agir efficacement en faveur du développement et pour la réparation de dangereuses décisions géopolitiques, comme en Libye par exemple ; pour mieux accueillir celles et ceux qui ne demandent pas l'aumône, qui ne viennent pas manger notre pain, mais nous demandent asile, aide, respect et dignité,

Le seul mot « immigration », tel le marteau du médecin sur le tendon rotulien, déclenche la phrase réflexe : « Vous faites le jeu du Front national. » Rassemblement national ! Les donneurs de leçons, qui aiment les mots pompeux, en ont trouvé un qui fait florès depuis quinze jours : il paraît qu'Emmanuel Macron « triangule Ils veulent dire par là qu'il braconne sur les terres des autres ... Je ne sais pas où il y a un triangle, mais passons. Quand les détenteurs du monopole du coeur comprendront-ils ce qui les a entraînés en salle de réanimation idéologique, l'angélisme et le victimisme, qui mettent les faits en fuite et qui, en déclarant tabous l'immigration et d'autres sujets, ont conduit les classes populaires à leur tourner les talons, comme on abandonne un matelas usé devant sa porte Le réel ne cessant pas d'exister parce qu'on l'ignore, on laisse à l'extrême droite le champ libre pour propager, avec une fixité de poteau indicateur, ses absurdités montées sur des échasses et ses pulsions xénophobes. Nous en avons eu un exemple tout à l'heure. C'est ainsi que les populistes sont aujourd'hui aux portes du pouvoir. Je ne vois donc pas de raison de me mêler au choeur des pleureuses : je vais parler de la politique migratoire et de l'intégration. Bien sûr, ce débat n'est pas sans risque. risque. Les deux bouts de l'omelette, comme disait Alain Juppé, sont en embuscade : il s'agit là d'un premier danger. « Ouvrez les frontières ! » contre « immigration zéro ! » : les fonds de commerce du gauchisme irresponsable et de l'extrême droite intolérante, deux rhinocéros au cuir épais, à la vue basse et toujours prêts à charger vont ressurgir. L'opposition républicaine, à gauche comme à droite, sera tentée de pimenter ses discours d'un peu de cette radicalité. Je voudrais inviter à y renoncer. Voilà quarante ans que l'immigration est l'exemple même de l'impuissance publique ans que nous faisons ce que dénonçait Richelieu, lequel disait : « Faire des lois et ne pas les faire exécuter, c'est autoriser ce qu'on veut interdire. » Cette phrase doit nous inciter à l'humilité.

Ils ne veulent plus voir à la télévision des réfugiés noyés et échoués sur les plages après avoir été abandonnés par les passeurs. Ils ne veulent plus voir les pays européens se livrer à des querelles de cour d'école chaque fois qu'arrive un bateau de migrants. Ils ne veulent plus voir Calais et Vintimille. Ils ne veulent plus voir les centaines de tentes alignées le long des boulevards et des quais. Ils ne veulent plus voir les prostituées albanaises ou africaines, esclaves tragiques de mafias dont on avait cru notre pays débarrassé à jamais. Au bois de Vincennes ! Ce que veulent les Français, c'est d'abord comprendre. Ils voient bien que le maintien des illégaux sur le territoire est un fléau pour les sans-papiers eux-mêmes, forcés à la précarité et à la clandestinité, et une épreuve pour la population, contrainte de voisiner avec les squats ou les ghettos. Ils souhaitent donc que les reconduites à la frontière soient effectives. Les Français ont compris que le sujet est non pas seulement national, mais européen. Néanmoins, ils ne comprennent pas que l'Europe n'ait ni le mandat ni les moyens de le traiter. Frontex va voir ses effectifs passer de 2 000 à 10 000 agents : très bonne nouvelle- moins bonne quand on apprend que le chiffre de 10 000 sera atteint en 2027 ... Les Français veulent que l'on trouve des solutions pour faire cesser le détournement des procédures d'asile. Quand les deuxième et troisième nationalités par le nombre sont les Albanais et les Géorgiens, dont les pays sont considérés comme « sûrs », c'est le signe que, là aussi, les mafias et les passeurs ont mis la main sur le système. l'essentiel est ailleurs. Le Président de la République l'a parfaitement compris, mais le sujet est tellement inflammable qu'il a dû l'aborder, comme dirait Nietzsche, avec des pattes de colombe. Il l'appelle l'« insécurité culturelle ». En langage direct, cela veut dire la « crise de l'intégration ». Au début des années quatre-vingt sont apparus deux mouvements de jeunes antiracistes. Leurs buts étaient les mêmes, mais les méthodes les opposaient. Le premier, France Plus, d'Arezki Dahmani, avait pour mot d'ordre l'intégration républicaine. Son slogan était : « Nous voulons le droit à la ressemblance. Le second, SOS Racisme, proposait le multiculturalisme. Abreuvé de subventions, surmédiatisé par tous les relais du jacklanguisme triomphant, il fit une entrée fracassante dans le paysage politico-intellectuel. France Plus, privée de tout moyen, disparut. Au début des années 2000, un nouveau président de SOS Racisme, Malek Boutih, homme de gauche responsable, propose un virage à 180 degrés, s'oppose radicalement à ce qui était devenu le politiquement correct multiculturel, condamne le différentialisme et fait l'éloge de l'intégration républicaine. Mais le mal était fait, et Malek Boutih se trouve rapidement congédié. Le victimisme et le dolorisme sont devenus l'alpha et l'oméga du discours d'une certaine intelligentsia sur l'immigration, ... C'est vrai ! ... un discours qui, au prétexte d'atténuer le déracinement des immigrés, conduit à les laisser à la discrétion de leur communauté un discours qui, au nom de la tolérance, renonce à les protéger contre les abus de la tradition dont ils relèvent. C'est ainsi que la France est devenue un pays où montent chaque jour un peu plus le communautarisme et les discours anachroniques de l'indigénisme, de la racisation ou de l'islamo-gauchisme. Le défi de l'intégration est immense, comme l'indiquent les sondages récents selon lesquels 27 % des musulmans pensent que la charia est supérieure aux lois de la République française. Mais ce chiffre montre aussi que la grande majorité d'entre eux pense le contraire. Et les très nombreux exemples chez les enfants et les petits-enfants d'immigrés aux parcours scolaires et professionnels réussis- chacun d'entre nous en connaît autour de lui -apportent un démenti aux victimocrates, qui expliquent l'échec de l'intégration par les obstacles rencontrés. démenti est encore plus éclatant : celui des centaines de milliers de boat people asiatiques, arrivés eux aussi dans les années quatre-vingt, sans connaître un mot de notre langue. Dès la deuxième génération, ils ont atteint le niveau moyen d'études et de revenu des Français. Leur chance, si l'on peut dire, c'est que notre modèle, ils en avaient rêvé pendant des années, contre la tyrannie qu'ils fuyaient par tous les moyens, comme ils me le disaient lorsque, président de Médecins sans frontières, je travaillais dans les camps de réfugiés du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

ces derniers ont été assimilés rapidement, c'est aussi parce que la France était sûre de son modèle républicain, de sa conception de la laïcité, de sa façon de vivre ensemble et de sa place dans le monde. Le plus grand défi aujourd'hui n'est-il pas de réussir l'intégration dans un pays qui voit ces valeurs s'estomper, comme s'efface peu à peu, à la surface de la mer, un visage de sable ? Le plus grand défi n'est-il pas de convaincre Français comme immigrés que ces valeurs sont non seulement celles du passé, mais aussi celles de l'avenir ? Cette question n'est pas posée qu'à vous, monsieur le Premier ministre, elle est posée à chacun d'entre nous. Elle est posée à notre démocratie

mon groupe écartent tout déni et se veulent force de proposition pour combattre le sentiment d'impuissance de l'État en matière de droit d'asile et de migrations. Ce sujet touche à l'essentiel, à la souveraineté et donc à l'État,

Notre ligne directrice sera de considérer que la modération des idées n'écarte pas la fermeté de l'action, et qu'en particulier en matière de droit d'asile un « non » doit être un « non », un « oui » doit être un « oui « oui ». Dans cet exercice contraint, je me concentrerai sur nos propositions. Notre première proposition porte sur la construction d'un droit européen de l'asile convergent. Monsieur le Premier ministre, vous nous l'avez dit, Entre le niveau le plus bas d'harmonisation- un soutien logistique, financier et technique par le bureau européen d'appui -et le niveau le plus haut- une harmonisation totale, avec une agence européenne de l'asile et un droit 100 % européen, en l'état, est un voeu pieux -, nous suggérons deux solutions. La première, qui a notre préférence, serait une coopération dite « renforcée » avec neuf pays au minimum, une sorte de premier cercle

sur une reconnaissance mutuelle des décisions prises quant aux demandes d'asile. Elle permettrait à ceux qui veulent avancer de le faire. La seconde solution, plus modeste, serait de travailler à la convergence par la technique, par des définitions communes des critères d'asile, ou encore par des référentiels partagés relatifs aux niveaux de risques dans les pays d'origine. L'élaboration de ces référentiels pourrait être confiée à un organisme européen de l'asile. Elle permettrait de converger vers une culture commune de la pratique du droit d'asile. En résumé, il s'agirait d'une convergence, faute d'unification.

appel au précédent. Mais, dans une décision du 14 mai 1996, la Cour constitutionnelle fédérale a élargi considérablement la notion de pays tiers sûr, ... C'est vrai ! ... en énonçant que « quiconque arrive d'un pays tiers sûr n'a pas besoin de la protection, car il aurait pu trouver une protection contre les persécutions politiques dans le troisième État ». C'est exactement ce que ne permet pas notre droit constitutionnel. Bref, les

mais le caractère essentiel de ce travail d'interopérabilité, couplé à une histoire informatique française qui a pu avoir ses défaillances, me conduit à vous suggérer une maîtrise d'ouvrage particulièrement robuste dédiée à cette mission

Nous sommes ouverts à l'idée, déjà débattue au Sénat, suivant laquelle le rejet de la demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, vaudrait OQTF, à la manière

la non-coopération des pays d'origine qui pose un problème majeur et la politique de réciprocité les conditions d'octroi des visas qui a ses limites. Cette question peut être traitée sous forme bilatérale- l'Espagne fait mieux que nous, par exemple, avec le Maroc -ou à l'échelon européen, en s'appuyant sur la conditionnalité des aides au développement. Cette mesure serait efficace si elle était couplée à

Nous serions favorables à l'idée d'un débat annuel devant le Parlement avec des orientations, voire des objectifs chiffrés, dont l'administration pourrait rendre compte en cas de non-réalisation. Nous sommes également ouverts à l'idée d'un statut de migrant temporaire avec permis de séjour et de travail, à la manière d'une européenne, assez similaire à l'autorisation temporaire pour les métiers en tension

Mon groupe est favorable à une analyse ciblée des conditions de résidence, de ressources, d'intensité des liens familiaux, ou encore de durée, sans pour autant remettre en cause les principes. Septième proposition : nous souhaitons la simplification des régimes d'hébergement.

suggestion concerne la question du travail. Un demandeur d'asile ne peut envisager de travailler avant un délai de six mois- neuf mois précédemment ; nous serions prêts à examiner l'abandon pur et simple de ce délai,

aux éternelles difficultés françaises des silos de décision, avec des sujets qui ne relèvent que du ministère de l'intérieur,

Je sais très bien qu'il serait injuste de vous rendre coupable de tous les échecs en matière de politique migratoire, mais en politique, on est toujours comptable de ses choix et de ses décisions.

Les chocs migratoires que nous avons connus il y a deux ou trois ans ne sont que les prémices de secousses telluriques beaucoup plus violentes qui se produiront lorsque l'Europe aura perdu, à la fin du siècle, 100 millions d'habitants alors que l'Afrique en aura gagné près de 2 milliards. Auguste Comte disait : « la démographie, c'est le destin

d'autres encore ont vu dans chaque homme un individu interchangeable et dans chaque migrant une ressource économique bon marché déplaçable et corvéable à merci.

lorsqu'il parle d'embourgeoisement et évoque le risque d'une société française coupée en deux, avec des catégories supérieures éduquées qui ont les moyens de se mettre à l'abri des effets de l'immigration par des stratégies d'évitement résidentiel et scolaire

indiqué que vous étiez prêt à corréler une politique humanitaire de développement de l'Afrique avec un effort, par ces pays

nous avons trop reculé, sur la laïcité, par exemple. Monsieur le Premier ministre, avez-vous renoncé à modifier la loi 1905 ? Nous devons tenir coûte que coûte et l'on voit bien que l'attentat à la préfecture de police nous appelle à cette résistance, chaque jour. Nous avons reculé sur l'assimilation. Regardons les choses en face : les valeurs républicaines d'égalité, de liberté, de laïcité, de fraternité civique, on les assimile, on ne les intègre pas.

généreuse de devenir complètement français. Mes chers collègues, relevons la tête, soyons fiers de nos convictions, ne cédons rien, parce que les Français nous le reprocheraient. Oui, la générosité fait partie du patrimoine, de l'héritage français, mais encore faut-il avoir quelque chose à donner, une histoire à offrir, des valeurs communes à partager, un pays à aimer. Rien ne serait pire, parce qu'il serait inhumain, qu'un monde sans frontières, où, de déracinements en affrontements, on dresserait les populations les unes contre les autres. Monsieur le Premier ministre, si vous souhaitez que ce débat ne soit pas seulement un signe d'habileté politique,

Après les interventions des orateurs des groupes, la parole est à M. le Premier ministre.

Sans surprise, je constate- nous l'avons tous entendu -que la question de la définition et de la mise en oeuvre d'une politique migratoire dans notre pays n'appelle pas, dans cet hémicycle, comme dans celui de l'Assemblée nationale, un consensus. Au fond, personne n'en est complètement surpris : entre les positions qui ont été développées par Mme la présidente

d'asile -et une certaine forme de fermeté, c'est-à-dire la capacité de choisir et de ne pas se voir imposer qui a le droit de résider sur le territoire national. Dans cette tension, difficile à mettre en oeuvre,

des positions nationales en Europe, ou la nécessaire construction d'une politique européenne était indispensable, s'agissant du contrôle des flux migratoires et de l'harmonisation, de la fluidification et de l'efficacité d'une véritable politique d'asile. Nous le sentons tous. Beaucoup d'entre vous ont présenté l'asile comme une question centrale au sein de la politique migratoire. En la matière, nous devons utiliser les pistes qui sont à notre disposition et prendre des initiatives diplomatiques en Europe

On dit souvent, en se tournant vers le passé, qu'elle était plus simple lorsqu'il s'agissait d'une immigration issue de

Le « modèle républicain » n'était pas si stabilisé au moment où les Italiens ou les Polonais sont arrivés en masse dans notre pays. Leur conception de la pratique religieuse était souvent bien différente de celle qui prévalait en France. Ces difficultés ont donné lieu à des violences, à des discriminations,

que l'Albanie est à un niveau de préparation justifiant le début des négociations avec l'Union européenne pour une éventuelle adhésion. De deux choses l'une

Je n'ai pas inventé ces procédures, mais je les ai mises en oeuvre quand j'étais maire. Il y a là comme un hiatus. Nous pouvons peut-être y travailler, je dis bien peut-être, parce que je ne suis pas sûr que nous trouvions la bonne solution, et surtout, je ne suis pas sûr qu'elle soit immédiatement efficace.

Troisièmement, quels seront les textes ou les supports des décisions à mettre en oeuvre ? Nous ne sommes pas venus dans ce débat annoncer un grand texte général qui serait la grande loi ou le grand soir législatif de la politique migratoire, traitant tous les sujets, depuis la relation diplomatique avec les pays d'origine jusqu'au retour vers les pays d'origine, ou jusqu'à l'intégration ou la citoyenneté.

d'accompagnement au développement des pays d'origine, et peut-être d'accompagnement des États dans la mise en place d'instruments qui leur seront utiles, ainsi

séance est reprise. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour une mise au point au sujet de votes.

Deuxièmement, cet amendement vise à faire de la conférence des maires une véritable instance de concertation en accordant à chacun de ses membres un droit de veto suspensif. Quel est l'avis de la commission ? Notre l'avis de la commission ? Notre collègue souhaite en premier lieu que les maires puissent être représentés éventuellement par un membre du conseil municipal à la conférence des maires de l'EPCI.

Je vous propose d'y intégrer également les maires délégués des communes nouvelles. En effet, la création de communes déléguées est très prisée au sein des communes nouvelles. Selon l'étude d'impact, seules 22 communes nouvelles sur les 239 créées au 1 janvier 2019 n'ont pas conservé des communes déléguées.

Il s'agit d'une réunion préalable à la réunion de l'assemblée délibérante, afin de recueillir l'avis des maires au sein de la conférence des maires sur les projets de délibération inscrits à l'ordre du jour. L'amendement a pour pour objet d'associer davantage le maire aux travaux de l'intercommunalité, mais aussi de garantir une meilleure prise en compte de l'avis des maires sur les délibérations du conseil communautaire, afin de recentrer les travaux de l'EPCI sur les besoins des communes.

Il s'agit d'une précision qui a été adoptée lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale. Grand, est ainsi libellé : La parole est à M. Jean-Pierre Grand. La création de la conférence des maires est obligatoire pour les métropoles et, si au moins 30 % des maires des communes membres en font la demande, pour les autres EPCI. La conférence des maires se réunit sur l'initiative du président de l'EPCI ou à la demande d'un tiers des maires.

comme c'est le cas pour les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants. Il est évidemment souhaitable que les maires soient informés avant de discuter des sujets au sein de la conférence des maires. Toutefois,

diversité des demandes montre l'hétérogénéité de la volonté des élus. Il est déjà prévu que la conférence des maires, si elle n'est pas créée par le pacte de gouvernance, puisqu'elle est

entre maires, et uniquement entre maires. Au-delà de ce calendrier qui pourrait être fixé de façon quasi rituelle sur l'ensemble de la durée du mandat, nous

Et tous les mois, elle était utile, non pas pour aborder les délibérations à venir du conseil communautaire, mais pour anticiper souvent très en amont les orientations futures et échanger avec l'ensemble des maires, ce qui permettait à l'administration de préparer des délibérations qui conviennent aux communes.

si par hasard le président de l'EPCI est récalcitrant, une sauvegarde existe. Donc, de grâce, n'en rajoutons pas ! Je m'inscris dans la logique qui a été exprimée par le Gouvernement. Essayons de donner un tout petit peu de souplesse ! Je trouve étonnant qu'au Sénat, alors que nous défendons les libertés locales, nous passions autant de temps à débattre de la manière dont les élus doivent faire leur boulot ! Avons-nous oublié, mes chers collègues, qu'avant la loi qui interdisait le cumul des mandats, nous avons tous été maire ou président d'EPCI. Si nous ne l'avions pas oublié, nous ne passerions pas autant de temps à nous demander comment les maires et les présidents d'EPCI doivent s'organiser.

Les maires des petites communes ont un sentiment d'inutilité au sein des intercommunalités. Ils sont parfois démotivés et participent peu ou pas aux choix de gouvernance. Leurs problématiques ne sont pas ou peu prises en compte, car elles ne sont pas identifiées comme d'intérêt communautaire. Il y va pourtant de la cohésion de l'ensemble intercommunal et du développement de projets pour tous. Pour recréer le sens et la cohésion nécessaires au territoire, il convient de donner la parole et les moyens d'agir aux élus de ces petites communes afin que l'intercommunalité ne se résume pas à la juxtaposition des projets de quelques maires ou communes très influents. Quel

la conférence des maires et le pacte de gouvernance sont justement faits pour répondre à cette nécessité d'entendre les maires de toutes les communes, quelles qu'elles soient. En effet, je vous rappelle que la conférence des maires fonctionne sur le principe «

dans chaque EPT de la métropole du Grand Paris sur le modèle de celle prévue pour les EPCI à fiscalité propre nous semble être une bonne idée. La commission émet donc un avis favorable.